séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie

texte. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que le texte qui nous réunit aujourd'hui parvienne au terme de son parcours parlementaire, à l'issue d'une commission mixte paritaire conclusive, dans une version équilibrée qui reprend très largement les apports du Sénat introduits lors de son examen en février dernier. Nous avions alors accueilli favorablement ce texte, qui offrira au secteur public un nouvel outil pour relever l'immense défi que représente la transition énergétique des bâtiments publics, soumis par la loi à d'ambitieuses obligations de performance énergétique. de ces travaux est estimé à 500 milliards d'euros pour l'ensemble du secteur public, à mobiliser d'ici à 2050. Fidèles à notre rôle constitutionnel de représentants des collectivités territoriales, il nous est par conséquent apparu nécessaire d'accompagner ces dernières dans la réalisation de ces travaux, favorisant ainsi l'atteinte des objectifs de performance énergétique que leur impose la loi. La solution prévue par ce texte peut représenter une avancée et permettre de débloquer de nombreux projets locaux : les acheteurs publics pourront plus facilement programmer des travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments, en faisant partiellement reposer leur financement sur les économies d'énergie qui résulteront de ces travaux, le coût initial étant pris en charge par un tiers-financeur. Il s'agit ainsi d'une dérogation au code de la commande publique, lequel prohibe, à juste titre, tant les dérapages sont possibles, le paiement différé. C'est pourquoi nous sommes restés attachés au principe d'une expérimentation, qui prendra fin au bout de cinq ans. Nous avons renforcé les exigences de suivi et d'évaluation de cette dernière, afin de nous assurer que les dérogations au code soient limitées, que les collectivités territoriales soient accompagnées et que soit ainsi évité tout accident financier. Sur ce point, nous avons accentué les conditions de soutenabilité financière des projets, conscients que le tiers-financement représente un coût final plus élevé pour l'acheteur public, le tiers-financeur répercutant son avance de trésorerie lors du paiement différé. Comme j'ai pu l'exprimer à plusieurs reprises lors des diverses étapes de la navette parlementaire, ce texte ne constituera pas une solution miracle effaçant les difficultés du secteur public en matière de rénovation énergétique. Il s'agit d'une solution complémentaire, certes bienvenue, mais qui ne nous dédouanera pas d'une réflexion d'ensemble sur les moyens de mettre en oeuvre la transition environnementale à l'échelon local. Nous serons donc attentifs à l'application qui sera faite de cette nouvelle faculté laissée aux mains du secteur public, en formulant le voeu que l'évaluation demandée par la loi que nous nous apprêtons à voter soit effective. Tous les apports du Sénat ont été maintenus lors de la commission mixte paritaire (CMP). C'est donc un texte presque identique à celui que nous avions adopté en février dernier qu'il vous est proposé de voter aujourd'hui. Outre des modifications rédactionnelles, la CMP a notamment permis d'inclure l'étude préalable parmi les documents transmis aux assemblées délibérantes devant approuver la signature du contrat- une précision utile -, et d'encadrer la durée du marché, celui-ci devant se limiter à la durée de l'amortissement des investissements. Compte tenu de ces avancées et du compromis qui a été trouvé, à l'unanimité, en commission mixte paritaire, je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de ce texte, qui permettra de trouver des solutions locales pour améliorer le quotidien des usagers du service public et respecter nos engagements en matière de décarbonation. La

parue hier, nous rappelle l'urgence d'agir face au réchauffement climatique, d'accélérer notre transition et, en particulier, d'avancer sur la décarbonation de nos sociétés. Ce défi majeur de la transition écologique passe nécessairement par la décarbonation des bâtiments, qui produisent 23 % des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Ce chantier crucial de la rénovation de nos bâtiments, nous l'avons déjà lancé, et il a un coût, notamment pour l'État et les collectivités dont le bâti représente 30 % du parc tertiaire national, avec un important potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique. C'est un chantier où l'État comme les collectivités se doivent d'être exemplaires. En effet, avec 75 % du parc des bâtiments publics, les collectivités territoriales sont tout particulièrement en première ligne. première ligne. Cette proposition de loi, qui vise à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique, parvient aujourd'hui au terme de son parcours parlementaire. Elle est à présent soumise à votre approbation.

Je tiens à saluer l'esprit dans lequel cette proposition de loi a été conçue, dans le dialogue avec les collectivités territoriales, les élus locaux et le Parlement, en particulier avec l'apport décisif du Sénat. Le texte a été débattu, enrichi, amendé, et cette version issue de la commission mixte paritaire est un bel exemple de compromis en vue de l'intérêt général. La qualité des échanges doit beaucoup aux rapporteurs, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et je tiens, madame la sénatrice Eustache-Brinio, à vous remercier personnellement de votre engagement. Le tiers-financement n'est ni une réforme du code de la commande publique- nous sommes dans une logique d'identification des bonnes pratiques et d'expérimentation -ni un désengagement de l'État. C'est une arme supplémentaire, mise à la disposition des élus qui le souhaiteront. Elle

Mesdames, messieurs les sénateurs, le chantier de rénovation du bâti public est une priorité de la lutte que nous menons contre le réchauffement climatique. Mais il n'y a pas, d'un côté, la question environnementale, et, de l'autre, les questions économiques et sociales. C'est le dernier point sur lequel je souhaiterais insister : la rénovation du bâti public a un coût, mais elle ouvre des perspectives extrêmement concrètes de réduction des dépenses. Investir pour rénover, c'est agir directement pour les finances de sa commune et de sa collectivité. Mais c'est aussi améliorer la vie de nos concitoyens, des agents qui travaillent dans ces bâtiments et de tous leurs usagers. Le texte qui vous est soumis est un texte de consensus, qui permettra de renforcer notre action publique pour le bénéfice de nos concitoyens, sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Il favorisera également la mobilisation de l'ensemble des acteurs du bâtiment, au service de la décarbonation du secteur, et leur ouvrira de nouvelles perspectives économiques sans lesquelles ce chantier systémique ne pourrait être mené à bien. C'est pourquoi je ne doute pas que l'adoption de ce texte fera l'objet d'un large consensus sur vos travées. Nous passons

on le sait, les dépenses en fluides représentent une part importante du budget de nos collectivités, surtout dans un contexte marqué par une crise de l'énergie couplée à une inflation galopante. Les bâtiments publics qui font la force et l'image de notre service public dans nos territoires doivent répondre aux enjeux du développement durable. Ils représentent près de 400 millions de mètres carrés, dont les trois quarts relèvent de la compétence directe des collectivités territoriales. Chaque année, l'énergie pour chauffer des équipements ou des bâtiments représente 2,6 % de la consommation finale d'énergie du pays.

Nous reconnaissons volontiers que cette proposition de loi semble un outil adapté pour accompagner la rénovation énergétique, notamment pour permettre à des communes, surtout dans les secteurs ruraux, de lever les freins à certains investissements. Lors de la commission mixte paritaire, les sujets sur lesquels nous avions eu des réticences et des interrogations n'ont pas été débattus : je pense notamment aux dépenses nécessaires et indispensables pour la mise aux normes des réseaux électriques, la sécurité, les systèmes anti-incendie, ou encore les normes

Madame la rapporteure, vous l'avez rappelé, lors de la commission paritaire mixte, notre abstention était bienveillante. Nous réitérons ce vote : le groupe CRCE s'abstiendra sur cette proposition de loi.

Nous nous félicitons que la CMP soit parvenue à un accord et que sa version soit presque identique à celle qui a été adoptée par le Sénat le 16 février dernier. Nous avions alors voté en faveur de ce texte à l'unanimité, exception faite de l'abstention, tout de même bienveillante, de nos collègues du groupe communiste

suppose de dégager pas moins de 400 milliards d'euros d'ici à 2050. Le défi est considérable. Il nous faudra mobiliser des ressources supplémentaires en quantité pour accomplir nos desseins en matière climatique, mais aussi pour améliorer les conditions d'accueil des usagers et des agents du service public, et, ainsi, réduire les factures énergétiques des collectivités, en particulier celles qui sont relatives aux bâtiments scolaires. Nul besoin de vous rappeler, mes chers collègues, l'ensemble des problèmes de financement auxquels sont confrontées les collectivités.

Il permettra de faciliter l'accès aux financements aux collectivités, à l'État et à leurs établissements en faisant partiellement reposer les investissements sur les économies d'énergie qui résulteront des travaux de rénovation, le coût initial étant pris en charge par un tiers-financeur. Concernant le texte en lui-même, cinq articles restaient en discussion et, comme l'a souligné Mme la rapporteure, outre des modifications rédactionnelles, la version que nous examinons maintenant ne diverge de celle du Sénat que sur des points mineurs.

Nous soutenons cette idée, car c'est une solution pertinente, d'autant qu'elle consiste en une expérimentation, ce qui nous permettra de procéder à une évaluation rigoureuse, puis, éventuellement, d'en corriger les défauts.

en faveur de la transition énergétique. Vous l'aurez compris, nous voterons en faveur des conclusions de la CMP sur ce texte. La parole

cette proposition de loi, qui devrait bientôt être adoptée définitivement, arrive à un moment particulièrement opportun, ce qui peut justifier cette nouvelle dérogation aux règles habituelles de la commande publique. En effet, les crises auxquelles l'État et les collectivités doivent faire face sont multiples.

Les bâtiments publics y contribuent en grande partie, puisqu'ils représentent 37 % du parc tertiaire national. Leur rénovation énergétique doit donc faire figure de priorité si le pays veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Elle doit aussi permettre aux Français de mieux vivre, dans un pays soumis, comme jamais auparavant, aux aléas climatiques, notamment à des canicules répétées. Cet objectif ambitieux doit être soutenu par des actions concrètes, dès aujourd'hui, et la rénovation thermique en est l'un des piliers. crise est géopolitique. La guerre en Ukraine a fait grimper à des niveaux vertigineux le coût des énergies. Elle remet en question notre modèle d'approvisionnement, et rend plus impérative encore la nécessité de réduire cette dépendance énergétique que nous payons si cher.

alors que le bâtiment est responsable de 76 % de la consommation énergétique des communes, les travaux de rénovation sont trop peu mis en oeuvre dans le secteur public, probablement parce que le coût d'investissement est trop élevé. il faudrait dépenser la somme colossale de 500 milliards d'euros d'ici à 2050 pour respecter les obligations de la loi en matière de rénovation énergétique. Cette somme est évidemment impossible à mobiliser pour l'État et pour les collectivités. de ce texte, de lever l'obstacle financier lié à l'investissement à consentir pour financer la rénovation des bâtiments publics. L'accord trouvé en CMP ne diffère presque pas du texte voté au Sénat, qui avait semblé satisfaisant, au point qu'aucun groupe n'avait voté contre. La proposition de loi vise donc à autoriser l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements au recours au tiers-financement pour des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, ils pourraient faire financer par un tiers un programme de changement d'équipement ou une rénovation de bâtiment. L'opération était jusqu'à présent impossible du fait des règles de la commande publique, qui interdisent tout paiement différé. Avec le tiers-financement, une fois les travaux terminés, la collectivité reverse au tiers-financeur une forme de loyer dont le montant équivaut aux économies d'énergie consécutives aux équipements installés, sur une période déterminée. Ce mode de financement pourrait permettre aux administrations de réaliser des travaux d'envergure, dont le coût serait lissé dans le temps. Si nous accueillons toujours favorablement les mesures de simplicité et d'efficacité, nous sommes également vigilants quand il s'agit d'assouplir les règles d'utilisation de l'argent public. Il ne faudrait pas, notamment pour des collectivités dont les finances sont déjà exsangues, contribuer à l'émergence de mauvaises pratiques ou de mauvaises dettes. La proposition de loi semble répondre à cette inquiétude. D'une part, il est prévu que l'expérimentation se limite à cinq ans ; correctement évaluée, elle nous permettra de voir si ce nouvel outil a été pris en main et s'il n'a pas entraîné de difficultés inattendues. D'autre part, un contrôle accru, notamment avec l'étude de soutenabilité, permettra d'identifier clairement les incidences budgétaires pour chacune des parties prenantes. Pour conclure, l'accord trouvé en CMP nous offre un compromis satisfaisant et retient l'essentiel des apports du Sénat. Le texte qui ressortira de notre examen répondra à un devoir d'exemplarité de l'État et des collectivités, à l'heure où l'on en demande beaucoup aux Français pour s'adapter, voire survivre aux différentes crises que j'ai mentionnées plus tôt. Il contribuera à l'atteinte des objectifs ambitieux que la France s'est fixés, tout en améliorant les conditions d'accueil des usagers et les conditions de travail des agents. Enfin, il permettra de réduire les factures d'énergie de l'État et des collectivités

Cette politique de réduction de l'empreinte carbone nationale concerne tout particulièrement les collectivités, qui possèdent une bonne partie des 400 millions de mètres carrés du bâti public. Dans de nombreuses communes, notamment rurales, ce foncier est aussi abondant que vieillissant. Pis, dans un contexte de hausse rapide des prix de l'énergie et de tensions budgétaires, effectuer des rénovations d'une telle ampleur est devenu à la fois plus nécessaire et plus délicat. Les auditions menées par la commission ont d'ailleurs révélé l'ampleur de la problématique, la direction de l'immobilier de l'État (DIE) allant jusqu'à estimer que, sans mobiliser des ressources supplémentaires dédiées, il ne sera pas possible d'atteindre les cibles En parallèle, les limites des outils juridiques disponibles sont rapidement devenues manifestes. Les signatures de contrats de performance énergétique (CPE) demeurent rares, sous la forme tant d'un marché global de performance que d'un marché de partenariat de performance

Il était donc indispensable d'apporter une réponse. Par conséquent, le Sénat a accueilli favorablement la proposition de loi de nos collègues députés et l'a utilement enrichie suivant les préconisations de notre rapporteure, Mme Eustache-Brinio, dont je salue la qualité du travail. Toutefois, comme elle l'a souligné à plusieurs reprises, les possibilités offertes par le recours au tiers-financement résultant de la proposition de loi doivent conserver une dimension strictement complémentaire. La politique de rénovation énergétique ne doit pas se limiter à une recherche de fonds privés, sans quoi elle risquerait de contribuer à fragiliser les finances publiques locales. Ce n'est clairement pas ce que nous souhaitons en assouplissant certaines limites imposées à ces mécanismes de financement. Pour cette raison, l'évaluation préalable du recours aux marchés globaux de performance énergétique et l'anticipation de leur soutenabilité budgétaire ont particulièrement retenu notre attention. Loin de dénaturer le texte initial, ces préoccupations nous ont permis de construire un texte plus solide. Face à la convergence d'intentions des députés et des sénateurs autour de ces objectifs, la commission mixte paritaire est parvenue sans difficulté à un accord sur un texte commun. Celui-ci reprend les apports du Sénat, comme l'extension du bénéfice du dispositif aux EPCI et aux syndicats d'énergie, ou encore la transparence renforcée sur les conséquences financières du recours au marché global de performance. Le compromis obtenu avec le rapporteur de l'Assemblée nationale sur les dispositions relatives à l'analyse de l'intérêt économique effectuée dans l'étude préalable nous semble satisfaisant. De même, l'ajout en CMP d'un alinéa prévoyant la prise en compte de la « durée d'amortissement des investissements » dans la durée du marché global de performance constitue un apport opportun, qui va dans le sens des remarques formulées au Sénat. Avant de conclure, je tiens à souligner que, cette proposition de loi créant un dispositif expérimental, il conviendra de mener une évaluation soigneuse, aussi bien après trois ans, par le biais du rapport prévu à l'article 2, qu'au terme de l'expérimentation, dans cinq ans. Ces évaluations seront essentielles, non seulement pour juger de l'efficacité de la future loi et de ses conséquences potentielles sur la situation financière des acheteurs publics, mais aussi pour observer les progrès effectués dans le sens de la réalisation des objectifs nationaux en matière de performance énergétique. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera en faveur de la proposition de loi, dans sa rédaction résultant des travaux de la CMP. La parole est à M. Dany Wattebled,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que la commission mixte paritaire soit parvenue à une rédaction commune sur l'ensemble des dispositions restant en discussion de cette proposition de loi.

Cette expérimentation représente une avancée majeure, que je salue. Adopté le 19 janvier dernier à l'Assemblée nationale, puis le 16 février suivant au Sénat, le texte a bénéficié d'apports constructifs de la part des deux chambres. Au fil des débats, le dispositif a gagné en souplesse et en simplicité. Il en a résulté un outil facilitateur, dont je suis certain que nos élus sauront tirer profit. Je suis particulièrement heureux que la commission mixte paritaire ait conservé une très grande partie des enrichissements proposés lors des débats au Sénat ; je pense notamment aux dispositions visant à améliorer la transparence sur les engagements financiers. Il est essentiel de pouvoir anticiper de manière précise les conséquences financières des engagements qui seront pris au travers de ce dispositif. Ces contrats sont bien encadrés et favoriseront l'accomplissement des projets de territoire défendus par nos élus, avec toutes les précautions qui s'imposent, afin d'aller vers une réduction importante de l'empreinte carbone dans les années à venir. Le Gouvernement remettra un rapport d'évaluation qui permettra une analyse rigoureuse du dispositif. Nous jugeons cela utile et serons particulièrement attentifs à l'étude de ses bénéficiaires, mais aussi à la nature des projets accompagnés,

dans nos territoires, à l'image de la sécheresse dramatique qui sévit en ce moment même dans de nombreux départements. Tous les outils en faveur de la transition écologique mis à la disposition de nos élus sont les bienvenus. Comme nous l'avons rappelé lors de l'examen du texte, cette expérimentation est un atout supplémentaire dans le jeu des élus locaux. Il est très important de leur faire confiance. Nous pouvons donc nous féliciter de participer ensemble à la création d'une nouvelle pratique vertueuse, qui s'ajoutera au panel des

Elle se pose aussi pour nos collectivités. Le Sénat, chambre des territoires, connaît bien les problèmes auxquels elles sont confrontées. La crise énergétique et les discussions sur le filet de sécurité ont montré que ces difficultés étaient présentes partout, en milieu rural comme en milieu urbain, dans les petites collectivités comme dans les grandes. Pour autant, les bâtiments publics sont loin d'être épargnés par la surconsommation d'énergie. Ceux de l'État et des collectivités locales sont responsables de 76 % de la consommation énergétique j'avais rappelé que la Cour des comptes, à l'automne dernier, avait noté l'incohérence et le risque d'inefficacité des mesures gouvernementales destinées à améliorer l'empreinte environnementale des bâtiments : « Le secteur du bâtiment, résidentiel et tertiaire, constitue en France la première source de consommation d'énergie. La politique de rénovation énergétique des bâtiments, à laquelle l'État a consacré plusieurs réformes législatives au cours de la dernière décennie, est un outil majeur pour la mise en oeuvre de la stratégie bas-carbone et l'accentuation de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre.

Le coût de la dette climatique est bien trop nocif pour notre société, et les dépenses énergétiques indues grèvent les finances publiques, en particulier les finances locales. On retrouve donc bien, dans le cadre du patrimoine public, la double peine que vivent les foyers, ce cercle vicieux que nous connaissons trop bien : le renoncement aux travaux de rénovation pour des raisons financières maintient des dépenses énergétiques abyssales. L'urgence est là ! Ce texte issu de la CMP est une première étape dans la gestion du coût très élevé de travaux souvent nécessaires a pour objet une expérimentation pendant cinq ans de l'aménagement du droit de la commande publique, particulièrement en matière de paiement différé. Conscient de l'attente des collectivités, et favorable à l'accélération de la transition énergétique des bâtiments publics, notre groupe est favorable à cette expérimentation, mais il continuera à exprimer sa prudence envers un risque de captation par le secteur privé d'une grande partie de la rentabilité des activités économiques suscitées par les économies d'énergie, à la faveur d'une forme de privatisation de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux et de leur financement. les fameux partenariats public-privé (PPP) ont souvent été accompagnés d'abus de la part des partenaires privés. L'inertie des dernières décennies a déjà un coût. Il convient de s'assurer qu'il ne soit pas encore amplifié. Au-delà de cette expérimentation, c'est bien la question du financement de la transition énergétique qui se pose, et je salue le constat de notre rapporteure à ce sujet : cette proposition de loi ne représente qu'« un dispositif complémentaire bienvenu, mais qui ne peut représenter l'unique solution pour réussir la transition énergétique du secteur public », d'autant que « le tiers-financement [ ...] ne doit pas être favorisé de façon systématique en raison des surcoûts finaux qu'il entraîne ». J'espère que beaucoup sur ces travées sont en accord avec le principe de pollueur-payeur et qu'ils défendraient ainsi une taxation des entreprises les plus polluantes pour mieux alimenter le budget de MaPrimeRenov'ou de tout autre dispositif d'aide à la rénovation des logements des particuliers

L'objectif de réduction de 60 % de la consommation énergétique des bâtiments publics d'ici à 2050 ne peut être atteint sans des mécanismes d'accompagnement, de préférence pérennes, lisibles et peu coûteux.

Nous en sommes loin. Une grande stratégie de rénovation thermique aurait dû et devrait être une priorité majeure de l'État, au même titre que notre stratégie énergétique. Néanmoins, ce texte va dans le bon sens. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera en sa faveur, en restant attentif aux dérives des marchés de rénovation.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, déposée le 29 novembre 2022 par les membres du groupe Renaissance, cette proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale le 19 janvier puis par le Sénat le 16 février suivant. Cette quasi-unanimité parlementaire a débouché, logiquement, sur une commission mixte paritaire conclusive, il y a deux semaines. Je remercie les deux rapporteurs, la sénatrice Eustache-Brinio et le député Cazenave, de leurs travaux. En moins de quatre mois, le Parlement se sera prononcé en faveur de l'ouverture du tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales, traduisant une volonté de soutenir la réalisation de travaux de rénovation énergétique. faut bel et bien accélérer, alors que la loi Élan a imposé en 2018 une réduction de 60 % de la consommation d'énergie finale des bâtiments publics d'ici à 2050 par rapport à leur niveau de 2010.

Il rend impératif un effort massif et continu, notamment budgétaire, afin de rendre possible la rénovation énergétique des 400 millions de mètres carrés concernés. L'objectif est triple : réduire nos émissions de CO2 et préserver notre environnement, diminuer les factures énergétiques à la charge de l'État et des collectivités territoriales, enfin, améliorer les conditions de travail des agents et d'accueil du public. C'est dans ce cadre d'action que le groupe RDPI a souhaité créer une mission d'information sur « Le bâti scolaire à l'épreuve de la transition puisque 12 millions d'élèves sont scolarisés chaque année. Face aux défis colossaux qu'il nous faut relever, de nombreux leviers doivent être activés, afin de bénéficier d'expertises juridiques et techniques de qualité, mais aussi pour faciliter et de diversifier les sources et les modalités de financement. Le dispositif innovant dont nous discutons aujourd'hui se veut une réponse pertinente pour ce faire. Il vient encourager et faciliter le recours des personnes publiques aux contrats de performance énergétique, qui sont encore trop peu utilisés. En levant quelques freins à l'investissement qui résultent du coût élevé que représentent les travaux, le texte que nous nous apprêtons à adopter définitivement vient déroger, sous forme expérimentale et pour une durée de cinq ans, au code de la commande publique. Il vise ainsi à engager plus facilement des travaux de rénovation énergétique en différant leur paiement. Il s'agit ni plus ni moins de lisser le coût de la rénovation en faisant porter par un tiers le paiement immédiat des travaux, d'où le terme de « tiers-financement ». Cela permettra un remboursement progressif, sous forme de loyer annuel, en partie réalisé grâce aux économies d'énergie induites.

mais qui, en matière de rénovation énergétique, ne sont presque jamais utilisés par les collectivités territoriales, et, d'autre part, aux marchés globaux de performance. Pour les élus locaux, le tiers-financement permettra de conserver la maîtrise d'ouvrage et de contractualiser en se qui intégrera le financement et la réalisation des travaux de bout en bout. Le texte de compromis trouvé en CMP ne diverge ne diverge du texte établi par le Sénat que sur quelques points mineurs, comme vous nous l'avez précisé, madame la rapporteure. En ce qui concerne l'article 1 , l'étude préalable à l'engagement de la procédure de passation d'un marché global de performance

Il a également été précisé que la durée du marché global sera déterminée « en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues » ; encore une fois, nous y sommes favorables. Le groupe RDPI votera pour ce nouvel outil mis au service de la transition énergétique. La parole

reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis heureuse de vous présenter les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à renforcer l'équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, alimentation saine, durable et accessible à tous. Le législateur tente de nouveau dans ce texte de réguler des relations commerciales plus tendues que jamais entre industriels et distributeurs, dans un contexte d'inflation croissante. Je me réjouis que nous soyons parvenus à un accord entre sénateurs et députés sur des points cruciaux, comme le rééquilibrage des rapports de force entre ces acteurs, en affirmant le caractère d'ordre public de notre droit commercial et en protégeant la valeur des matières premières agricoles, donc le revenu des agriculteurs. Les discussions ont été vives, compte tenu des éléments nouveaux que le Sénat a introduits dans le texte et des divergences de vues initiales entre nos deux assemblées, notamment sur les articles 2 et 3, mais nous avons su trouver des compromis au service de l'intérêt général. Je tiens à souligner l'écoute et la qualité des échanges sur ce texte, que ce soit entre nous, mes chers collègues, ou avec l'auteur et rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, M. Frédéric Descrozaille- qu'il en soit remercié, ainsi que ses équipes. ses équipes. La grande majorité des apports du Sénat, et ils sont nombreux, ont été conservés par la commission mixte paritaire. Premièrement, nous avons contribué à protéger l'emploi, l'investissement et l'innovation dans nos territoires, en mettant fin pour les

Deuxièmement, nous avons complété le dispositif de protection des matières premières agricoles au sein des négociations commerciales, pour une plus juste rémunération des agriculteurs. En effet, si ces matières premières sont sanctuarisées pour ce qui est de la négociation sur les marques nationales ce n'était pas le cas pour les produits vendus sous marque de distributeur (MDD), alors même que ces produits prennent de plus en plus de place dans les rayons. C'est désormais chose faite. Dans la même perspective de protection des filières agricoles, la commission mixte paritaire a conservé l'exclusion de la filière des fruits et légumes du dispositif

Depuis 2018, le Sénat pointe la fragilité de ce dispositif opaque, unique en Europe, qui consiste à donner un chèque en blanc aux distributeurs en espérant qu'ils utiliseront cette marge pour mieux rémunérer les producteurs. En CMP, nous sommes tombés d'accord avec nos collègues députés pour exercer un contrôle renforcé et raccourcir d'un an la durée de l'expérimentation, jusqu'en 2025. Quatrièmement, les avancées du Sénat sur les pénalités logistiques ont été conservées. Si leur existence même n'est pas contestable, encore faut-il qu'elles soient utilisées à leur juste mesure et à bon escient par les distributeurs. Les dispositions que nous avons adoptées permettront de s'en assurer.

Le compromis trouvé permet seulement au fournisseur, à titre expérimental, de choisir entre cesser subitement de livrer ou appliquer un préavis de rupture qui tiendra compte des conditions économiques du marché.

Cette proposition de loi, sur laquelle le Sénat va se prononcer définitivement, contribuera à la poursuite du rééquilibrage des relations commerciales dans la chaîne agroalimentaire et, ce faisant, à un meilleur partage de la valeur au bénéfice des agriculteurs.

À cet égard, ce texte va globalement dans le bon sens, en particulier sur la nécessaire prolongation du dispositif expérimental de relèvement du seuil de revente à perte de 10 % pour les produits agricoles et alimentaires. Cette prolongation constituait une attente très forte du monde agricole. Sur ce point, j'aimerais saluer ici l'esprit d'ouverture dans lequel les travaux du Sénat ont été conduits. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale proposait de prolonger l'expérimentation jusqu'en 2026. C'était aussi, vous le savez, la position exprimée clairement par le Gouvernement. En commission, le Sénat a manifesté ses doutes- ceux-ci sont toujours utiles -à l'égard de ce mécanisme, qu'il a proposé de le suspendre durant deux ans, le temps que la période inflationniste que nous traversons prenne fin. J'avais alors rappelé devant vous, à l'occasion de l'examen du texte, qu'il s'agissait non pas d'opposer le revenu des agriculteurs à la protection du pouvoir d'achat des ménages, en particulier les plus modestes, mais bien de mener ces deux combats de front. J'avais rappelé qu'il fallait, à mon sens, assumer collectivement le fait qu'une alimentation de qualité, sûre, produite dans des conditions respectueuses de notre environnement et de notre biodiversité ait un coût. le maintien d'un outil de production agricole et agroalimentaire dans nos territoires avait un coût. Et j'avais constaté avec vous que l'évaluation de cette expérimentation avait été rendue difficile par la crise sanitaire, à laquelle avait succédé un choc inflationniste concomitant de la guerre en Ukraine. Il semblait donc nécessaire au Gouvernement de prolonger cette expérimentation, mais avec les dispositifs de contrôle et d'évaluation adéquats, pour répondre aux préoccupations légitimes de votre commission et de votre rapporteur.

Bien sûr, le Gouvernement demeure convaincu qu'une prolongation de trois années à périmètre constant aurait été plus adaptée en termes de lisibilité et de cohérence du dispositif pour les acteurs des relations commerciales. Je pense naturellement à la désynchronisation des dates entre encadrements des promotions et SRP+10, ainsi qu'à l'exclusion des fruits et légumes sans justification préalable. Toutefois, malgré ces deux réserves, l'équilibre global auquel la CMP est parvenue me semble satisfaisant. J'en viens maintenant à l'article 3, qui fixe les modalités de la relation commerciale entre fournisseurs et distributeurs en cas d'échec de la négociation annuelle. Cette disposition, très discutée, avait pour objectif d'apporter une réponse adaptée à un angle mort des négociations commerciales annuelles. Les opérateurs, qu'ils soient fournisseurs ou distributeurs, ont un intérêt commun à ce que les flux de ventes ne s'interrompent pas en cas d'échec de la négociation annuelle. Mais la relation commerciale doit parfois s'interrompre. C'est précisément cette situation qui requérait un encadrement juridique beaucoup plus précis.

L'écriture retenue en CMP laisse un choix clair au fournisseur et dispose que tout préavis tient compte des conditions économiques de marché, précision ô combien utile en période inflationniste. Par ailleurs, le recours à la médiation pour conclure un préavis est facultatif, ce qui évitera l'engorgement des saisines du médiateur et le report systématique que nous pouvions craindre de la date butoir. C'est un texte qui a atteint son point d'équilibre en évitant les écueils que les versions antérieures avaient pu soulever. C'est aussi un texte empreint d'une certaine prudence, parce qu'il est expérimental. L'apport décisif du Sénat sur cet article doit être salué. Je salue également le rehaussement des amendes administratives pouvant être infligées en cas de non-respect de la date du 1 mars. Je serai attentif à ce que nos services de contrôle s'en saisissent pleinement, afin de lutter contre les pratiques de certains distributeurs tentés de jouer la montre pour mettre la pression sur les producteurs. Permettez-moi d'être moins disert sur les autres avancées de cette proposition de loi, que le Sénat a contribué largement à améliorer. Le souhait d'un encadrement renforcé des pénalités logistiques est exaucé, avec des obligations plus précises et des sanctions alourdies. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez veillé au caractère opérationnel de cet enrichissement de notre cadre législatif. Il faut en finir avec cette exception très française consistant de la part de certains acteurs à reconstituer leurs marges par l'application de pénalités abusives. Le mécanisme de suspension de l'application des pénalités logistiques en cas de circonstances exceptionnelles est également tout tout à fait pertinent. En témoignent les crises d'ampleur traversées ces dernières années, comme celle du covid-19, qui viennent légitimer auprès de nos concitoyens l'usage par l'État de ce type de prérogative régalienne. Par ailleurs, la proposition de loi consacre la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve des dispositions applicables du droit de l'Union européenne, pour connaître des litiges portant sur les négociations commerciales annuelles. Il s'agissait d'un autre angle mort de notre droit qu'il convenait de rectifier. Comme vous, le Gouvernement a particulièrement à coeur de lutter contre les comportements de contournement de la loi française que nous constations tous. Le texte apporte enfin quelques correctifs bienvenus à la loi Égalim 2, notamment en ce qui concerne la clause de renégociation, le fonctionnement de l'option 3

des produits alimentaires entre les mois de février 2022 et février 2023 selon l'Insee. Au-delà d'un mois de mars alarmant, c'est la preuve qu'une année noire vient de s'écouler pour les Français. Cette inflation inédite des prix de l'alimentation frappe en premier lieu les portefeuilles des consommateurs les plus modestes, ce que nous ne pouvons accepter. Notre action en faveur du pouvoir d'achat ne signifie pas pour autant que nous devons pénaliser les petites et moyennes entreprises, les coopératives agricoles et nos exploitations qui font tout pour que les Français puissent bénéficier de produits de qualité au prix le plus compétitif possible. Pour ce faire, nous devions corriger le déséquilibre inhérent à la relation fournisseurs-distributeurs, qui demeure très souvent défavorable à nos producteurs.

Nous pouvons aujourd'hui nous féliciter d'avoir conservé les principales avancées du Sénat dans la rédaction finale. Je pense tout d'abord à l'ancrage définitif du principe de non-négociabilité des matières premières agricoles et de sa déclinaison pour les produits vendus sous marque de distributeurs.

de ces exploitations étaient réels. Enfin, nous avons fait un pas en avant non négligeable concernant l'encadrement de l'arme absolue des distributeurs : les pénalités logistiques. Les dérives et les excès étaient connus.

Le plafonnement du montant des pénalités logistiques et le renforcement de leur encadrement sont de véritables victoires pour l'ensemble de ces industriels et de ces exploitations agricoles qui assurent l'approvisionnement des Français au quotidien. En sus de ces avancées, je me réjouis de voir que la commission mixte paritaire a su trouver un compromis concernant l'encadrement de la période de négociation commerciale annuelle. En cas d'échec de ces négociations, l'alternative proposée entre l'interruption des livraisons et l'application du préavis de rupture « classique » constitue un consensus

Parce que cette proposition de loi est un texte exigeant, qui met en lumière certaines limites du droit en vigueur, et parce qu'elle est le fruit d'un travail de compromis avec l'ensemble des acteurs politiques, économiques et des mondes

La CMP a été conclusive, et nous devons nous en réjouir, car le contexte de négociations commerciales tendues, dans une période d'inflation galopante, qui induit des efforts communs, Mais les efforts sont-ils communs ? L'inflation, qui fait la une de tous les médias, nous assène des hausses de prix incroyables : 14 % pour l'alimentation et jusqu'à 30 % pour la viande dans certains endroits. Le trimestre du panier anti-inflation a commencé par un constat mitigé de la part des consommateurs, ceux d'entre eux qui vivent dans la précarité ne pouvant acheter les produits dont les tarifs ont pourtant baissé. Dans cette guerre des prix, les distributeurs s'achètent une conscience tout autant qu'une image en affichant un objectif bienveillant : faire supporter le moins possible au consommateur les Mais qui paye ? On parle d'un financement grâce à la baisse des marges. C'est oublier que la guerre des prix a toujours été à charge pour les producteurs. Et ce sont les agriculteurs, une fois de plus,

La France, bon élève, en haut du tableau d'honneur, perd en compétitivité : quand le bio, par exemple, se vend au prix du conventionnel, un énorme problème se pose, qu'il faut résoudre rapidement.

la LME, qui a permis à la grande distribution de mutualiser la mise en place de centrales d'achats. Cette mesure a renforcé la pression sur les agriculteurs. Nous devons y travailler et tirer,, un bilan objectif après quinze Dans ce contexte commercial tendu, toute mesure positive pour les agriculteurs doit être encouragée et défendue. Mon groupe salue donc plusieurs avancées. L'article 1, tout d'abord, rappelle que les dispositions du code de commerce s'appliquent à toute relation contractuelle dès lors que les produits que celle-ci vise sont commercialisés en France. Il s'agit ici de contrer le phénomène d'évasion juridique consistant à délocaliser la négociation contractuelle, afin de la soumettre à des dispositions juridiques plus favorables et moins protectrices des intérêts des agriculteurs français et du fabriqué en France.

L'exclusion de la filière des fruits et légumes du dispositif est maintenue, conformément à plusieurs amendements adoptés par le Sénat, notamment celui de ma collègue Nathalie Delattre. La CMP a conservé la disposition introduite par le Sénat sur la non-négociabilité des matières premières agricoles des produits vendus sous marques de distributeur. C'est à mon sens C'est à mon sens un acquis important. Un grand pas est également franchi avec l'expérimentation de rupture des livraisons en cas d'échec des négociations commerciales annuelles entre un fournisseur et un distributeur. Cette mesure répond clairement à un enjeu d'équilibre entre ces deux parties. Je salue Mme la rapporteure, Anne-Catherine Loisier, qui a déclaré : « Le Parlement est obligé d'intervenir, non pas par plaisir, mais parce que les acteurs se livrent à une partie de " poker menteur " qui se fait souvent au détriment des consommateurs, des agriculteurs et des PME. » Vous avez bien raison, la rapporteure, et nous sommes nombreux à partager ce constat. Toutefois, ne soyons pas trop naïfs, car cela pourrait se retourner contre les agriculteurs français, la concurrence mondiale étant à l'affût. Dans une économie de marché libérale qui se conjugue à un contexte d'inflation exacerbée, les distributeurs achèteront ailleurs. L'article 1 est donc fondamental pour enrayer ce risque. Bref, la voie est bonne, mais il faut persévérer, car l'un des problèmes majeurs de notre agriculture est le faible revenu. Alors que se profilent le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricoles, le sujet du prix rémunérateur doit être l'un des enjeux primordiaux de notre réflexion.

que nous nous penchons sur un texte visant à réglementer les relations entre agriculteurs, producteurs, transformateurs, industriels, fournisseurs et distributeurs. Si nous y revenons, c'est non pas par coquetterie, mais par nécessité.

Derrière ces questions se pose celle de notre capacité à rester l'une des premières puissances agricoles et celle de notre souveraineté alimentaire, donc le problème central de notre indépendance.

Nous saluons les avancées trouvées en commission mixte paritaire, qui reprennent des apports importants du Sénat. Depuis la loi Égalim 1, nous sommes tous animés par le même objectif : faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, du fournisseur au consommateur, en passant par le distributeur. Nous le savons, l'équilibre n'est pas facile à trouver. L'article 2 relatif à l'expérimentation du seuil de revente à perte a fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause ! L'efficacité du dispositif n'a toujours pas été prouvée. La prolongation de l'expérimentation nous permettra, nous l'espérons, d'apporter des précisions.

L'autre avancée concerne l'exclusion des grossistes du système des pénalités logistiques. Nul ne conteste l'utilité des pénalités en cas de non-respect des obligations du contrat, qui permet de s'assurer que le distributeur sera bien livré dans les temps et conformément à ce qu'il a commandé. Cependant, des dérives ont été constatées. Les pénalités logistiques semblent être devenues une façon, pour la grande distribution, de compenser des pertes de marge sur certains produits. Ces dispositions ont donc été revues dans cette proposition de loi. Elles ont d'ailleurs été portées par plusieurs sénateurs du groupe Les Indépendants - République et Territoires, l'objectif étant d'éviter que les règles des pénalités logistiques n'aillent à l'encontre de la filière et de ses intérêts. l'article 3, il fallait régler le vide juridique existant lorsque fournisseurs et distributeurs ne trouvent pas d'accord et empêcher que, dans certains cas, un fournisseur ne puisse livrer à perte contre sa volonté. Depuis le début, la loi Égalim n'a pas apporté des résultats à la hauteur des espoirs suscités. C'est pourquoi nous y revenons pour proposer des améliorations. À n'en pas douter, nous y reviendrons encore. Nous en sommes à la saison 3 d'Égalim, et ce n'est sûrement pas la dernière de la série ! Même si nombre d'entre nous croient au marché, nous savons qu'il a besoin de règles, d'un cadre et d'un suivi, afin de nous assurer que, dans le prix final du produit payé par le consommateur, chaque acteur soit rémunéré à sa juste valeur. Monsieur le ministre, je le répète, nous attendons beaucoup de la future loi agricole. Nous sommes à vos côtés pour travailler sur les futurs pacte et loi d'orientation et d'avenir

l'inflation alimentaire poursuit sa course, avec pour conséquence des difficultés pour les producteurs, les fournisseurs et, bien sûr, un grand nombre de nos concitoyens. Dans ce contexte, nous nous apprêtons à voter une nouvelle loi pour tenter de rééquilibrer les rapports de force au sein de ces relations commerciales.

Si le texte que nous allons voter aujourd'hui comporte quelques avancées, on ne peut que douter de son efficacité, comme de celle des textes qui l'ont précédé. Certes, de petits pas sont effectués pour corriger les déséquilibres du système. Je pense notamment aux mesures sur les MDD, les pénalités logistiques ou la lutte contre les contournements de la loi les centrales étrangères. dans un secteur marqué par une forte opacité et des rapports de force violents, l'incertitude sur l'efficacité des mesures et leurs effets de bord éventuels persiste, comme le montre la question du seuil de revente à perte. En effet, si on peut se satisfaire

il faut des mesures bien plus structurantes pour trouver l'équation garantissant à la fois un revenu à nos agriculteurs et une accessibilité à une alimentation durable et de qualité pour tous. la première partie de l'équation, sans régulation des marchés, sans clauses miroirs, sans paiements pour services environnementaux, sans une PAC plus juste, sans une promotion du commerce équitable, nous ne parviendrons pas à rémunérer correctement les producteurs. Nous nous devons de sortir l'alimentation d'une concurrence mondiale délétère, qui est l'une des principales causes de la faiblesse du revenu agricole. Je voudrais ici évoquer l'accord avec le Mercosur, une nouvelle fois.

J'en viens maintenant aux consommateurs. Les mesures visant à mieux rémunérer les producteurs doivent s'accompagner de politiques fortes pour un accès à l'alimentation durable et de qualité pour tous, en particulier dans un contexte d'inflation.

et accès à l'alimentation durable. Nous continuons donc de plaider pour une véritable sécurité sociale de l'alimentation. Sans grand espoir, nous

la correction de dérives inadmissibles, qui sont le fruit du déséquilibre dans le rapport de force et dans les négociations commerciales. Il faut sans cesse s'adapter à la créativité d'un certain nombre de centrales-

Je me réjouis que le texte de la CMP maintienne les éléments essentiels de la proposition de loi initiale portée par Frédéric Descrozaille, ainsi que des ajouts issus du Sénat,

un bon équilibre. Cela permettra, à titre expérimental, que le fournisseur ait le choix entre l'interruption des livraisons, si le prix durant le préavis est jugé trop bas, ou l'application d'un préavis de rupture classique, qui devra tenir compte des conditions économiques du marché. Il s'agit d'un apport très intéressant de notre assemblée. Nous pouvons donc être fiers de parachever la protection du revenu agricole dans les négociations. Nous agissons pour préserver l'emploi, l'innovation et l'investissement dans nos territoires. Dans la presse Dans la presse quotidienne nationale, ces derniers jours, un distributeur a trouvé les moyens de publier des placards selon lesquels cette loi viserait à limiter les prix bas. Non, je le dis, cette loi vise à obtenir des prix justes,

Alphonse Karr, célèbre écrivain et journaliste français du XIXsiècle, écrivait : « En France, on parle quelquefois de l'agriculture, mais on n'y pense jamais.

Or qui sont les vraies victimes de l'inflation et de l'augmentation du coût des intrants et de l'énergie ? Sur qui se répercutent les hausses ? Sur les consommateurs, bien sûr, mais aussi sur les agriculteurs.

Mes chers collègues, à la veille d'une grande loi agricole que nous appelons de nos voeux, nous devons impérativement nous intéresser à la situation de nos agriculteurs. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs ! La situation n'est pas le seul fruit de la covid-19 ni de la guerre en Ukraine. Force est de le constater, la conjoncture n'est pas la seule responsable de ce manque de résultats. Égalim 1 et Égalim 2 n'ont pas fait leurs preuves. Nous sommes loin du compte, et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le groupe socialiste avait pourtant alerté le Gouvernement sur le manque d'ambition de ces textes au vu de la gravité de la situation de notre agriculture. En effet, la ferme France est en déclin, notre agriculture souffre. Pourtant, des solutions existent. Dans , Jean-Jacques Rousseau écrivait : « La condition naturelle à l'homme est de cultiver la terre et de vivre de ses fruits. Mes chers collègues, nous devons mener bataille pour assurer notre souveraineté alimentaire. Nous le savons, le juste partage de la valeur est la condition d'un modèle vertueux. Agriculteurs, transformateurs et distributeurs, tous doivent trouver leur compte dans les négociations commerciales. Nous déplorons que ce texte ne fasse pas de la question des agriculteurs le coeur de sa réflexion. Mais tel n'était sans doute pas son objectif Il s'agit d'une proposition de loi d'ajustement, qui, malgré ses lacunes, permet tout de même un certain nombre d'avancées que nous saluons. Tout d'abord, nous nous félicitons que la plupart des améliorations votées par le Sénat aient été conservées dans la version finale. Bien qu'ils aient des répercussions trop marginales sur les revenus des agriculteurs, nous sommes satisfaits du prolongement de l'expérimentation du SRP+10 et, surtout, de l'exclusion des fruits et légumes du dispositif. Mon groupe et moi-même avions notamment porté cette revendication de la filière par voie d'amendements. Nous saluons aussi la réaffirmation du principe de la non-négociabilité de la matière première agricole pour les produits vendus sous marque de distributeur.

la constitution de centrales d'achat à l'étranger, pour échapper aux règles encadrant les négociations commerciales, telles qu'elles sont issues des lois Égalim. N'en déplaise à la grande distribution, s'il y a des règles, c'est pour qu'elles soient respectées, et notre rôle est d'y veiller.

Le texte que nous votons aujourd'hui n'a pas pour vocation d'inverser la vapeur. Selon moi, il ne donnera pas une toute-puissance aux transformateurs. Il s'agit au contraire d'équilibrer une situation qui ne l'était pas. Forcément, il y a des mécontents.

à des prix abordables, quitte à rogner sur les marges de la distribution. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l'aurez compris, les socialistes voteront ce texte, même si nous considérons qu'il n'est qu'une goutte d'eau. Il doit s'inscrire dans une réforme globale de notre modèle agricole, dans le cadre d'une réflexion plus large à laquelle nous souhaitons être associés. Je souhaite qu'il permette un rééquilibrage des relations commerciales entre industriels et distributeurs, ce qui devrait avoir, par ruissellement, des répercussions sur les producteurs. La parole

du producteur au consommateur, de la fourche à la fourchette. Nous sommes invités à voter un texte dont l'objet affiché est de mieux protéger tous les acteurs de la filière, ce qui est fort louable du point de vue de l'intention, mais quasiment impossible dans le cadre dans lequel nous évoluons. Les produits alimentaires connaissent une hausse spectaculaire, les prix de l'énergie restent à la hausse et nos agriculteurs demeurent confrontés à cette difficulté structurelle découlant du fait que l'essentiel de la valeur ajoutée des produits alimentaires ne revient pas à la production. La vie chère s'installe de manière durable, et les salaires ne suivent pas. Au fond, consommateurs, salariés et paysans sont confrontés au même problème de la juste rémunération de leur travail. Nous assistons à une hausse des prix, dont on ne sait pas toujours exactement à quoi elle est due, à une croissance faible, à une inflation forte et à un système économique saturé. Et ce sont toujours les mêmes qui en font les frais proposition de loi n'était pas de traiter la question des salaires ni du retour de la valeur ajoutée à la ferme. Pourtant, dans l'agroalimentaire, la proportion des entreprises voulant relever leurs prix atteint 70 %, ce qui laisse augurer une poursuite de la flambée des prix. Le Gouvernement nous a annoncé la création prochaine d'un « chèque alimentaire pour les plus modestes », dont on ne connaît aucun détail. Nous savons seulement que le Gouvernement ne « souhaite pas distribuer d'aide alimentaire au niveau global, pour s'assurer que les consommateurs ne fassent que les consommateurs ne fassent pas le choix de la malbouffe dans les grandes surfaces. » Le pays est au bord de la rupture, il s'appauvrit, et nous continuons à débattre d'une proposition de loi qui ne résoudra malheureusement pas le problème.

Nous ne voulons pas décourager les bonnes intentions qui sous-tendent ce texte. Dans le même temps, nous en mesurons toutes les limites.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales (proposition n° 344, texte de la

commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, l'enfance a été placée par le Président de la République au nombre des priorités du nouveau quinquennat, et la protection des droits des enfants est au coeur de la feuille de route du Gouvernement qui en fait un engagement fort et prioritaire. « Le foyer familial doit être érigé en sanctuaire protecteur au sein duquel il ne saurait être accepté la moindre violence. » Voilà la directive ferme et sans ambiguïté que j'ai adressée à tous les procureurs de France dans ma dernière circulaire de politique pénale générale, en septembre dernier. Oui, la protection des mineurs exposés aux violences intrafamiliales est l'une des priorités absolues de ma politique pénale. Déjà, dans une circulaire du 21 avril 2022 relative à la prise en charge des mineurs présents lors d'un homicide commis au sein du couple, j'ai incité les procureurs à conclure localement des protocoles de prise en charge du traumatisme des mineurs présents lors d'un homicide commis au sein du couple, afin qu'ils soient accompagnés J'ai rappelé par circulaire du 28 février 2022 les dispositions du décret du 23 novembre 2021 énonçant que « lorsqu'un mineur assiste aux violences commises au sein du couple, il n'en est pas simplement le témoin, il en est victime à part entière ». Je demande ainsi aux magistrats de restituer aux faits commis en présence d'un mineur leur exacte qualification, de veiller à la préservation des droits du mineur dans la procédure pénale et de s'assurer que la juridiction de jugement dispose d'informations lui permettant de statuer sur l'autorité parentale. Je vous annonce la diffusion cette semaine d'une nouvelle circulaire de politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs. Cette circulaire porte la lutte contre les violences sur mineurs à un niveau équivalent à celui mis en oeuvre en matière de violences conjugales, dans la continuité des actions qui ont été menées ces dernières années. Porter cette politique ambitieuse et nécessaire implique de lutter non seulement contre toutes les formes de violences qui sont faites aux mineurs dans leur quotidien proche, qu'il s'agisse du cadre familial ou institutionnel- scolaire, parascolaire, sportif, culturel, religieux, etc. -, mais également contre toutes les formes d'exploitation, comme la prostitution, dont ils sont victimes, notamment de la part de réseaux organisés. Vous connaissez aussi ma volonté de généraliser les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger (Uaped), avec mes (Uaped), avec mes collègues François Braun et Charlotte Caubel, dont je veux saluer l'engagement. Je sais également pouvoir compter sur tous les juges des enfants, tous les juges aux affaires familiales (JAF) et tous les membres du parquet, qui exercent leurs missions au quotidien sur l'ensemble du territoire afin de protéger l'enfant dans son intégrité physique et morale, et de veiller à la préservation de ses intérêts. Enfin, je n'oublie évidemment pas votre engagement, celui du Sénat, dans ce domaine. En témoignent les textes que vous avez été nombreux à voter au cours de l'année écoulée. Car si le foyer familial doit être ce lieu de la sécurité affective, il est malheureusement des situations où il devient un lieu de persécution. Il en est ainsi lorsque l'un des parents devient le bourreau de l'enfant. Ces situations viennent bouleverser le présupposé naturel sur lequel repose la relation parent-enfant.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 Lorsque le parent maltraitant n'est à l'évidence plus en mesure d'assurer ce rôle, il faut nous résoudre à remettre en cause le lien parental. Ces questionnements ont été menés au cours de la précédente mandature lors des travaux parlementaires relatifs à la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Ils vous ont conduit à doter notre droit de dispositifs innovants à même de protéger l'enfant dans sa relation avec un parent maltraitant. Je pense, tout d'abord, au mécanisme de suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent qui est poursuivi ou condamné pour avoir commis un crime sur l'autre parent. Introduit à l'article 378-2 du code civil, c'est ce dispositif que l'article 1 de la présente proposition de loi vise à étendre. de la possibilité pour le juge pénal de retirer l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent qui a été condamné pour un crime ou un délit sur l'autre parent ou sur son enfant, objet de l'article 2 de la présente proposition de loi. Les débats que nous menons aujourd'hui démontrent toutefois que ces dispositifs peuvent et doivent encore être améliorés. À l'heure où l'ampleur du traumatisme engendré par les violences sexuelles n'est plus à démontrer, les conclusions intermédiaires de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants font ce constat alarmant qu'un adulte sur dix a été victime de violences sexuelles dans son enfance. Si l'enfance est le lieu privilégié des abus, il y a donc urgence à agir afin de s'assurer que le parent maltraitant ne puisse continuer à se prévaloir de ses droits pour maintenir une emprise sur son enfant ou pour réitérer ses agissements. L'Assemblée nationale- en particulier la députée Isabelle ainsi que les membres de la majorité -ne s'y est pas trompée lors de ses travaux, pas plus que votre commission des lois, en adoptant le texte que nous allons examiner aujourd'hui et qui vise à renforcer la protection de l'enfant victime de violences intrafamiliales. L'article 1 de la proposition de loi tend à modifier l'article 378-2 du code civil afin d'étendre Le texte adopté élargir le mécanisme de suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en cas de poursuite ou de condamnation du parent pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de l'enfant. La rédaction retenue par la commission des lois est opportune à bien des égards. Le choix de viser tous les crimes commis sur l'enfant constitue ainsi une amélioration sensible du dispositif puisqu'il évite d'introduire une hiérarchie inopportune entre les crimes dont un enfant peut être victime. Il le limite toutefois aux infractions les plus graves afin de garantir la constitutionnalité et la conventionnalité du dispositif. Une disposition miroir est prévue à l'article 2 de cette loi pour permettre une délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale dans ces hypothèses, initiative que je soutiens fortement. Il est cependant que la commission des lois n'ait pas repris le mécanisme qui, dans ces cas de suspension, dispensait le parquet de saisir pour une confirmation le juge aux affaires familiales, car on constate en pratique ce n'est que très rarement fait. Cette situation n'est d'ailleurs pas sans poser quelques difficultés quant au rétablissement ou non des droits de l'autre parent L'article 2 de la proposition de loi tel qu'il est issu des travaux de votre commission tend à créer trois mécanismes de retrait facultatif de l'autorité parentale ou de son exercice. la volonté de votre commission, madame la rapporteure, de renforcer la protection des enfants. Toutefois, cet article 2 ne permet pas d'atteindre pleinement cet objectif. En droit positif, le juge pénal a déjà l'obligation de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice en cas de viol, d'agression sexuelle ou de violence. Il apparaît plus efficace et et protecteur de l'intérêt de l'enfant de créer un mécanisme de retrait obligatoire de l'autorité parentale ou de son exercice pour les crimes et les agressions sexuelles incestueuses commis sur l'enfant et les crimes commis sur l'autre parent, avec une possibilité pour le juge d'y déroger par une motivation spéciale. Il s'agit là de mettre en oeuvre les recommandations du rapport intermédiaire de la Ciivise. L'article 3, quant à lui, vise à ne pas laisser le code pénal en reste et à le faire évoluer en conformité avec les modifications introduites dans le code civil. J'observe que la rédaction de cet article laisse transparaître un souci de simplification puisqu'il procède manifestement de la volonté d'inciter les magistrats à faire directement usage des dispositions du code civil, auquel il est renvoyé. l'intérêt de regrouper en un article unique du code pénal les dispositions qui ont trait à l'autorité parentale, lesquelles sont en droit positif dispersées dans différents chapitres du code pénal. En la matière, la simplification est évidemment la bienvenue. Je suis d'avis de parfaire cette idée en soutenant l'un des amendements visant à ajouter dans votre texte une expression

la commission a également souhaité introduire la possibilité, pour la juridiction de jugement, de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Je suis réservé quant à cette disposition, car elle porte en elle un risque, qui n'est pas à écarter, d'augmentation de la charge des audiences et, subséquemment, des délais d'audiencement, lesquels sont un facteur à part entière de l'efficacité de la justice. Il conviendrait que le texte précise bien qu'un tel renvoi de la décision portant sur l'autorité parentale ne peut intervenir qu'une fois la décision sur la peine Les réflexions doivent donc se poursuivre dans le cadre de vos débats. J'ai à coeur d'aboutir avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, à un dispositif ambitieux, ambitieux, mais respectueux de nos principes constitutionnels. Aussi, je forme le voeu que nos débats nous permettent d'envoyer un signal fort à tous les enfants victimes de violences intrafamiliales.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je me réjouis que le Gouvernement n'ait pas engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi d'Isabelle Santiago, ce qui nous permettra de travailler dans la durée sur un sujet éminemment complexe : la question de l'autorité parentale en cas de violences intrafamiliales. Je tiens aussi à féliciter notre vise à intervenir ponctuellement sur deux mécanismes : la suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale, créée par la loi du 28 décembre 2019, et le retrait de l'autorité parentale par les juridictions pénales.

comme le droit de consentir au mariage ou celui de consentir à l'adoption de son enfant. C'est donc la titularité même qui est mise en cause. Le retrait de l'exercice de l'autorité parentale revient, quant à lui, à confier exclusivement à l'autre parent le soin de veiller sur l'enfant et de prendre les décisions nécessaires pour sa santé, son éducation, etc. Pour autant, l'autre parent conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant les droits de visite et d'hébergement qui lui sont accordés, sauf « motifs graves » appréciés par le JAF. Il conserve aussi un droit de surveillance qui oblige l'autre parent à le tenir informé de tous les choix importants relatifs à la vie de l'enfant. Cela étant rappelé, venons-en à la proposition de loi dont nous sommes saisis. L'article 1 vise tout d'abord à étendre la suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement aux cas de poursuites ou de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant. La commission a été favorable à cette extension qui permet de prendre en compte la situation de l'enfant et non pas seulement celle de l'autre parent, se conformant ainsi aux souhaits de la Ciivise. L'article 1 tend également à revoir les conditions de durée : au lieu d'une durée maximale de six mois et d'une obligation pour le procureur de la République de saisir le JAF dans les huit jours, la suspension courrait jusqu'à la décision de non-lieu, la décision de la de la juridiction de jugement ou la décision du juge aux affaires familiales, s'il est saisi par le parent poursuivi. Sur cette question, la commission a choisi de s'en tenir à la position qu'elle avait adoptée en 2020 lorsqu'elle avait été saisie d'amendements similaires, similaires, en acceptant une suspension de plein droit, mais uniquement pour six mois, et en exigeant une intervention du juge pour la suite. Il nous semble en effet disproportionné, au regard de la présomption d'innocence et du droit de chacun de mener une vie familiale normale, de permettre une suspension automatique tout le temps de la procédure pénale, qui peut durer plusieurs années, et sans intervention obligatoire d'un juge, seul à même d'apprécier l'intérêt de l'enfant. Enfin, les députés ont créé un régime de suspension distinct en cas de condamnation pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours sur l'autre parent. Le texte vise à prévoir dans ce cas une suspension provisoire de l'autorité parentale, mais uniquement si l'enfant a assisté aux faits. La suspension vaudrait jusqu'à la décision du JAF, qui devrait être saisi par l'un des parents dans les six mois à compter de la décision pénale. À défaut, le parent retrouverait l'exercice de l'autorité parentale. ne nous a pas semblé cohérent à cause de la condition liée à la présence de l'enfant- car un enfant, même non présent au moment des violences, peut tout autant ressentir la souffrance et l'insécurité -, et à cause de l'exclusion des violences volontaires sur l'enfant lui-même. dispositif nous a semblé manquer d'intérêt pratique puisque les juridictions doivent d'ores et déjà se prononcer sur l'autorité parentale en cas de condamnation pour cette infraction. Je relève que les magistrats sont de plus en plus sensibilisés à l'importance des mesures relatives à l'autorité parentale et que le nombre de mesures prononcées augmente, ce dont on ne peut que se réjouir. L'article 2 de la proposition de loi vise ensuite à rendre plus « automatique », sans toutefois l'imposer au juge pénal, le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle commis sur l'enfant ou pour un crime commis sur l'autre parent. Cette disposition a le mérite d'inciter plus fortement les juges à prononcer un retrait total d'autorité parentale en cas d'infraction grave contre l'enfant ou l'autre parent, sans toutefois les priver de leur liberté de moduler leur décision au regard de l'intérêt de l'enfant, à charge pour eux de la motiver spécialement. La commission des lois en a revu la rédaction afin de rendre le dispositif plus intelligible, et donc d'en favoriser l'application par les juridictions pénales. Elle a posé le principe du retrait total de l'autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle commis sur l'enfant ou pour un crime commis sur l'autre parent, et l'obligation des juridictions de se prononcer dans tous les cas de condamnation d'un parent pour crime ou délit commis sur son enfant ou pour crime commis sur l'autre parent. Nous aurons tout à l'heure un débat sur cette rédaction : celle que nous avons choisie a le mérite de la vérité puisqu'elle expose clairement que le juge conserve malgré tout, sous réserve d'une motivation spéciale, la possibilité de ne pas prononcer le retrait total de l'autorité parentale. Les formules du type « prononce le retrait » ou « ordonne le retrait » nous semblent de ce point de vue relever davantage de l'affichage ... L'article 2 de la proposition de loi vise ensuite à ajouter un nouveau cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant par un parent qui est seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. La commission y a apporté un simple ajustement rédactionnel. La commission a adopté un article additionnel 2 pour pour instituer un « répit » pour l'enfant en cas de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement. Il tend à prévoir qu'aucune demande au juge aux affaires familiales ne puisse être présentée par le parent moins de six mois après le jugement. Une disposition similaire existe en cas de retrait de l'autorité parentale et il nous a semblé opportun de le prévoir aussi en matière d'exercice. J'en arrive à l'article 3, qui vise à procéder à diverses modifications dans le code pénal, à des fins de coordination avec l'article 2. Cet article nous a semblé l'occasion de mettre fin au décalage qui existe entre le code civil et le code pénal en matière de retrait de l'autorité parentale. La rédaction proposée introduirait une disposition générale dans le code pénal, applicable à chaque fois qu'il y a condamnation d'un parent pour crime ou délit sur la personne de son enfant ou l'autre parent. La commission s'est attachée à rendre les dispositions dont elle était saisie plus intelligibles et plus cohérentes, étant consciente qu'il fallait faciliter le travail des pénalistes pour qu'ils s'emparent de ces mécanismes de nature civile. C'est dans cet esprit constructif qu'elle a adopté le texte que je vous invite à voter. Nous avons besoin de bonnes lois, mais aussi d'une volonté politique absolue et de moyens dans les juridictions. C'est à ce prix que nous pourrons protéger les plus fragiles et infléchir ce monde de violence. Nous devons tous être des protecteurs de l'enfance et des guetteurs de violence. Car cette violence au sein de la famille empêche un enfant, tout simplement, de vivre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, c'est l'histoire de Malakai, un petit garçon âgé de 7 ans, battu à mort dans la nuit du 12 au 13 octobre 2022 par le compagnon de sa mère. Celui-ci avait déjà été condamné huit fois pour des faits de vols, de menaces et de violences conjugales. Pourtant, en avril 2022, les services sociaux s'étaient saisis du cas de la mère et de son fils, qui avaient fait l'objet d'un signalement à la justice en raison de « carences éducatives et de conduites addictives de la mère et d'un père totalement absent ». La mort tragique de Malakai est loin d'être anodine. En France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents dans un contexte de violences conjugales. À ce titre, 400 000 enfants vivent dans un foyer où s'exercent des violences conjugales et 160 000 enfants subissent chaque année des violences sexuelles. Les travailleurs sociaux croulent sous les dossiers qu'ils ne parviennent plus à traiter, faute de moyens suffisants. De surcroît, les tribunaux dénoncent une dégradation dramatique de la situation du pôle des affaires familiales. Les JAF sont débordés et en sous-effectif, mais je ne vous apprends ici rien de nouveau ... Dans tout ce désordre judiciaire, y a-t-il une place à à consacrer à l'intérêt supérieur de l'enfant ? La responsabilité de l'État est immense. Aujourd'hui, nous discutons d'un texte qui vise à améliorer la protection des enfants en renforçant le dispositif existant de retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Désormais, tout parent ayant été poursuivi, mis en examen ou condamné pour un crime commis sur l'autre parent et/ou crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant se verra suspendre de plein droit l'exercice de l'autorité parentale, ainsi que les droits de visite. Cette proposition de loi pourrait être une réelle avancée en matière pénale et civile. Certes, cela n'est toujours pas suffisant pour lutter contre les violences intrafamiliales. Le Gouvernement devrait élaborer une véritable politique publique ambitieuse en matière de protection de l'enfance. On ne peut pas se contenter de petites mesures ou de numéro vert. C'est notre devoir d'empêcher qu'un autre Malakai ne meure sous les coups d'un parent violent. Il nous faut garantir un accompagnement effectif pour tous ces enfants victimes de violences intrafamiliales

le groupe RDSE se réjouit de la présentation de cette proposition de loi, qui soulève des enjeux primordiaux et nous ramène à notre responsabilité collective de protéger nos enfants. Notre édifice institutionnel et législatif relatif à la protection des enfants doit s'enrichir de nos débats. Je rappelle que le groupe RDSE, sensible à la question de la protection des enfants, s'est déjà positionné sur un renforcement de la répression des abus sexuels intrafamiliaux. Les violences intrafamiliales sont le quotidien d'un trop grand nombre de nos concitoyens. Pire encore, celles dont sont victimes nos enfants posent un problème dont notre société a du mal à reconnaître le caractère massif et systémique.

Chocs traumatiques, troubles psychotraumatiques, phénomènes de dissociation, troubles de la mémoire : derrière ces violences, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, les conséquences sur l'enfant et son développement sont graves. Néanmoins, rappelons qu'elles sont réversibles si une protection et un traitement psychothérapique spécialisés sont mis en place. Nous plaidons pour une mise à l'abri rapide des enfants victimes et une prise en charge la plus précoce possible, afin de limiter les conséquences sur leur santé. Tout retard dans cette mise en sécurité et cette prise en charge équivaut à une perte de chance pour chaque enfant concerné. Au-delà des questions d'élargissement du mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et de systématisation du prononcé du retrait de l'autorité parentale par les juridictions pénales, notamment en cas de crime commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent ou d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant, nous devons nous interroger sur la bonne temporalité pour agir et protéger l'enfant en coupant le lien avec le parent violent, que ce soit de façon temporaire ou définitive. cette réflexion sans perdre de vue l'objectif de protection des victimes et de préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous devons également mettre l'accent sur une meilleure sensibilisation de la société sur ces sujets, afin de traiter le plus en amont possible les violences intrafamiliales sur la personne de l'enfant. Si la législation progresse depuis quelques années, il nous faut faire mieux, d'abord en accroissant l'arsenal législatif en matière de suspension et de suppression de l'autorité parentale ou de son exercice, sans oublier de rendre davantage lisibles et applicables les mesures déjà en place dans le droit en vigueur. Dans ce cadre, le groupe RDSE se félicite des avancées que comporte ce texte, notamment l'élargissement du régime de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement aux crimes et agressions sexuelles incestueuses commis sur la personne de son enfant. Cependant, nous regrettons que la commission ait souhaité atténuer la portée du dispositif principal en excluant la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale du parent violent le temps de la procédure pénale. Si cette modification répond au principe de présomption d'innocence et au droit de chacun, enfant comme parent, de mener une vie familiale normale, elle ne permet pas, compte tenu notamment de la longueur de la procédure pénale, d'améliorer un

Prévenir ou guérir ? Tel est le dilemme qu'affrontent les acteurs de la protection de l'enfance. Où doit-on placer le curseur ? Toujours est-il qu'il serait opportun que nous trouvions des solutions afin que notre appareil répressif ne souffre plus d'une ineffectivité dont les conséquences peuvent être lourdes. Néanmoins, en dehors de ces quelques observations, nous pensons que cette proposition de loi va dans le bon sens et contribuera à briser davantage le silence autour des violences commises dans le cadre intrafamilial. La systématisation du prononcé du retrait de l'autorité parentale par les juridictions pénales en cas de crime commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent ou d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant en est le formidable symbole. C'est pourquoi le groupe RDSE votera cette proposition de loi. La parole

le retrait de l'autorité parentale est, dans notre culture, encore difficile à envisager. Pourtant, cette option reste nécessaire dans l'éventail des moyens de protection de l'enfant victime de sa famille. Depuis des décennies, les philosophies des acteurs de la protection de l'enfant s'affrontent. Le législateur doit trancher : pour nous, il est indispensable de sanctionner le parent coupable de violences extrêmement graves sur l'enfant et de protéger cet être vulnérable physiquement en l'éloignant juridiquement de l'autorité dont il dépend et qui le détruit.

J'avais à l'époque remarqué que de nombreux enfants placés, en principe temporairement, étaient oubliés dans leur lieu de placement, sans surveillance, par l'administration toute puissante. Les enfants étaient souvent transférés à la campagne, au vert, loin des « mauvais parents ». Ceux-ci n'avaient plus de droits sur la vie de leurs enfants du fait, non de la loi, mais de la toute-puissance de l'administration.

Mais il n'abordait pas le devenir des enfants. La seule mesure pérenne pour eux était le placement, le plus souvent irréversible. La loi du 4 juin 1970 a remplacé la puissance paternelle par l'autorité parentale. Elle marque une étape essentielle dans l'évolution de la protection de l'enfant en ce qu'elle consacre l'égalité des parents. À partir de cette époque, si le magistrat peut retirer l'enfant de sa famille en cas de nécessité, il doit s'efforcer, par principe, de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et faire en sorte que les liens soient maintenus dans la mesure du possible. Le législateur de l'époque a cependant prévu une divisibilité des prérogatives de l'autorité parentale. La loi prévoit ainsi de diminuer les possibilités légales des père et mère quant à l'éducation de l'enfant si son intérêt le justifie. Le législateur présente les mesures restreignant l'autorité parentale en respectant une gradation. Les magistrats, dès lors, peuvent limiter, voire retirer, l'autorité parentale des parents. Cependant, dès cette époque, le législateur invite les juges à considérer la mesure prise comme provisoire et à recourir le plus souvent possible à l'assistance éducative. En ce qui concerne les mesures judiciaires propres à l'enfant, la loi du 6 janvier 1986 est venue renforcer les droits de la famille, en exigeant que les mesures soient limitées dans le temps, Aujourd'hui, la révision des situations est orientée avant tout vers le retour de l'enfant dans sa famille, quoi qu'il en soit. Avant les lois de décentralisation de 1983, la protection de l'enfant en danger reposait sur l'État. et à la protection de l'enfance qui a organisé la protection de l'enfance en danger. Cette loi fixe les attributions du département. Elle établit les responsabilités de prévention, de détection et de protection des enfants maltraités en redéfinissant le rôle de chaque

Je voterai ce texte, car il replace l'enfant victime au coeur du dispositif judiciaire. Coordonner le civil et et le pénal est une priorité pour la protection de l'enfant victime. C'est mon intime conviction. Le retrait de l'autorité parentale peut être nécessaire pour arrêter la reproduction de la violence familiale au sein des générations suivantes, mais il faut, en même temps,

Il provient d'une méta-analyse conduite par le Conseil de l'Europe, reprenant plusieurs estimations de diverses organisations indépendantes, comme l'Unicef ou l'OMS. Le rapport Sauvé, rendu public en octobre 2021, a donné une autre estimation, avec près de 15 % des femmes et plus de 6 % des hommes majeurs qui auraient été sexuellement agressés lorsqu'ils étaient mineurs. Cela ramène la prévalence dans la population totale à un peu plus de 10 %, comme l'a précisé M. le ministre. En tout état de cause, il s'agit d'un phénomène massif.

il est difficile de savoir si les violences sexuelles contre les enfants ont tendance à gagner du terrain, ou si nous en prenons davantage conscience à mesure que la parole se libère sur le sujet. Quoi qu'il en soit, il serait irresponsable d'ignorer ce phénomène qui brise les individus et divise les familles. En outre, les violences sexuelles ne sont qu'une partie du problème, sans doute la plus glaçante et la plus révoltante, mais une partie seulement. Les enfants subissent d'autres formes de violences au sein du foyer. En 2019, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes estimait à 400 000 le nombre des enfants concernés par ces violences. Il s'agit bien sûr des violences subies par les enfants eux-mêmes, le plus souvent à cause d'un père violent. Mais il s'agit aussi, et il ne faut pas le négliger, des violences qu'ils ne subissent pas directement, mais qui sont infligées par l'un des parents à l'autre. Celles-ci peuvent traumatiser les enfants presque autant que lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes d'éclats de colère, de coups ou d'insultes. Dans chacune de ces situations, la famille n'est plus le cocon protecteur qui permet à l'enfant de s'épanouir en sécurité ; la famille devient une prison dont il ne peut plus s'échapper.

C'était un préalable indispensable, car, en matière de violences intrafamiliales, une seule boussole doit guider l'action publique : l'intérêt de l'enfant. C'est pourquoi cette proposition de loi doit contribuer à faire avancer le débat sur ces sujets délicats et sensibles. Ils sont délicats, car il n'existe pas de solution miracle. Nous parlons de situations où l'agresseur est, par définition, un proche de la victime, et même le plus souvent un élément structurant de sa famille. Punir l'agresseur est nécessaire, mais parfois douloureux, malheureusement, pour la victime. Ces sujets sont également sensibles, car nous avons souvent, dans notre entourage, connaissance d'une situation particulière, d'un cas de figure où la violence a déjà assombri les relations familiales. Je rappelle au passage qu'il s'agit d'un phénomène qui dépasse tous les clivages sociaux et territoriaux. Je tiens à saluer Mme le rapporteur, qui a conduit un travail sérieux sur ce sujet complexe. Le texte de la commission nous paraît plus respectueux de l'intérêt de l'enfant, alors même qu'il peut paraître moins sévère contre les parents violents. Je le répète : notre seule boussole doit rester l'intérêt de l'enfant. plus précisément sur la réécriture de l'article 1. La commission a limité l'extension de la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale aux cas de crime ou d'agression sexuelle commis sur la personne de l'enfant. Elle a également souhaité conserver le caractère provisoire de cette suspension, comme c'est déjà le cas actuellement. Je le répète, il s'agit de sujets délicats et sensibles. En tant que législateurs, nous devons veiller à préserver la présomption d'innocence et les relations au sein des familles où sévissent de telles violences. C'est pourquoi il nous paraît judicieux de préserver aussi le rôle du juge aux affaires familiales dans l'application des sanctions à l'encontre des parents violents. Le législateur doit veiller à ne pas se substituer au juge. Rendre automatique le retrait de l'autorité parentale et de son exercice ne nous semble pas la réponse idoine.

Vogel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quand on ne peut pas se protéger soi-même, on doit pouvoir appeler à l'aide. Et quand on appelle à l'aide, on doit nous croire. Et quand on nous croit, on doit nous aider. Ces principes très simples devraient aller de soi. Pourtant, les protections accordées aux enfants victimes de violences intrafamiliales sont en France largement insuffisantes. Or il y a urgence, compte tenu de l'ampleur du phénomène : 165 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année ; 400 000 enfants vivent dans un foyer dont un membre exerce des violences conjugales, et en sont les victimes directes ou collatérales ; 2 enfants par classe et 1 à 2 adultes sur 10 ont été victimes de violences sexuelles, soit entre 35 et 70 d'entre nous, au Sénat, avec les fractures perpétuelles que cela implique. Les violences subies pendant l'enfance ont de graves conséquences psychologiques et somatiques qui durent souvent la vie entière. Le mouvement #MeTooInceste et la Ciivise, créée en réaction, ont démontré que la clé n'était pas tant la parole que l'écoute, car les victimes qui parlent ne sont que rarement crues, encore moins aidées convenablement, Il y a donc urgence à agir pour renforcer le cadre légal pour la protection des victimes. À cet égard, je remercie Mme Isabelle Santiago de son initiative et Mme la rapporteure, Marie Mercier, de son travail. L'ensemble du groupe écologiste soutient bien évidemment cette proposition de loi, qui est une étape importante pour améliorer la protection des victimes. En particulier, elle permettrait d'élargir les cas de suspension d'exercice de l'autorité parentale, afin de protéger l'enfant du parent violent. Si l'on croit la parole des victimes, il faut les protéger et, dans les cas de violences intrafamiliales, cela veut dire aussi parfois qu'il faut les protéger de leurs propres parents. C'est pourquoi l'élargissement de ces cas est une bonne chose. À ce titre, je voudrais m'attarder sur deux points qui me paraissent particulièrement importants. Premièrement, je regrette que la commission ait voulu supprimer certaines dispositions adoptées à l'Assemblée nationale. en particulier, de ne pas étendre la suspension de l'exercice de l'autorité parentale dans certains cas qui avaient été prévus par les députés. Or cette suspension est souvent essentielle pour permettre, dans les faits, la protection des enfants victimes de leurs parents violents. Le mouvement #MeTooInceste nous a montré que, dans de trop nombreux cas, on ne croit pas les victimes. Et comme on ne les croit pas, elles ne sont pas protégées par la justice. C'est ce que l'Assemblée nationale a retenu, et c'est pour cette raison que les députés ont voté pour un élargissement de cette suspension. Aussi avons-nous déposé des amendements visant à rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale.

Or, au lieu de protéger l'enfant en retirant l'exercice de l'autorité parentale, la justice remet parfois en cause le récit du parent protecteur et le suspecte d'accuser l'ex-conjoint pour se venger et d'instrumentaliser l'enfant.

chers collègues, 400 000 enfants vivent aujourd'hui dans un foyer où s'exercent des violences intrafamiliales, et un enfant en meurt tous les cinq jours. Par ailleurs, plus de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, selon un rapport de plusieurs inspections datant de 2018. Ces chiffres sont éloquents, ils sont d'une tout autre ampleur dans les territoires d'outre-mer. Dans une étude de 2017, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) rapportait que les violences intrafamiliales étaient plus fréquentes et plus graves outre-mer qu'en métropole, et ce en raison de l'insularité et de la faible superficie de certains territoires, qui peuvent entraver la libération de la parole et rendre inopérant l'éloignement du conjoint violent ou le choix d'un lieu anonyme pour être accueilli et écouté sans crainte.

L'un des enjeux de la lutte contre les violences intrafamiliales est de mieux reconnaître la souffrance des enfants qui en sont victimes et de les protéger. Nous savons aujourd'hui que les traumatismes répétés qu'ils subissent peuvent déclencher diverses maladies et être un facteur de reproduction de violences à l'âge adulte. Aussi, dans le prolongement du Grenelle des violences conjugales, lancé par le Gouvernement le 3 septembre 2019, le Parlement avait adopté deux lois prévoyant le renforcement des pouvoirs du juge pour retirer l'autorité parentale ou son exercice au parent violent, et pour protéger l'enfant et le parent victime. Tout d'abord, la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a notamment créé un mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a, entre autres dispositions, ajouté les délits commis sur l'autre parent à la liste des infractions pouvant fonder une décision de retrait de l'autorité parentale par le juge pénal. Pour traiter ces violences, notre arsenal juridique s'est, certes, considérablement renforcé ces dernières années, mais il reste encore perfectible.

et prévoit la mise en place de mécanismes automatiques de retrait ou de suspension de l'autorité parentale, ou de son exercice, lorsque le parent est poursuivi, mis en examen ou condamné pour les infractions les plus graves commises sur son enfant ou sur l'autre parent. Depuis son dépôt, des modifications substantielles ont été apportées au texte, toujours dans un esprit transpartisan et dans le cadre d'un travail de coconstruction avec le Gouvernement, qui a fait de la protection des mineurs exposés aux violences intrafamiliales une priorité absolue de sa politique pénale. Entièrement réécrite par l'Assemblée nationale, qui l'a adoptée à l'unanimité, cette proposition de loi prévoyait plus précisément d'élargir les cas de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement premièrement, jusqu'à la décision du JAF éventuellement saisi par le parent poursuivi ou jusqu'à la décision de non-lieu ou la décision de la juridiction de jugement en cas de poursuite, mise en examen ou condamnation pour un crime commis sur l'autre parent, ou de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant ; deuxièmement, jusqu'à la décision du JAF qui devrait être saisi par l'un des parents dans les six mois à compter de la décision pénale en cas de condamnation, même non définitive, pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits. La proposition de loi prévoyait également le retrait systématique de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur l'enfant ou pour crime sur l'autre parent, sauf si le juge en décidait autrement, à charge pour lui de motiver spécialement ce choix. Par ailleurs, elle ajoutait un nouveau cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant par un parent, seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Sur l'initiative de notre rapporteur, Marie Mercier, dont je tiens à souligner la qualité du travail, notre commission a choisi de réserver le déclenchement du mécanisme de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement aux crimes et agressions sexuelles incestueuses commis sur la personne de l'enfant. Nous approuvons cette position, mais il nous semble indispensable de prévoir le retrait de plein droit de l'autorité parentale ou de son exercice et des droits de visite et d'hébergement en cas de condamnation d'un parent pour ce même type d'infraction commise sur son enfant ou pour un crime commis sur l'autre parent. Nous vous présenterons, au cours de la discussion, trois amendements visant à concrétiser le plus fidèlement possible les recommandations de la Ciivise et à sécuriser la portée du dispositif. Au-delà de ces aménagements qui, je l'espère, recueilleront votre assentiment, nous débattrons dans les heures qui viennent d'un texte équilibré, tenant compte de la nécessité de protéger l'enfant et de préserver les relations familiales et des liens d'attachement. Voilà pourquoi le groupe RDPI, que je représente, votera en faveur de son adoption.

c'est une bien triste litanie que je reprends : près de 400 000 enfants en France vivent dans un foyer où des violences intrafamiliales sévissent ; dans 21 % des cas, ils en sont directement victimes. Ces violences- nous le soulignons tous -leur laissent des séquelles psychologiques et physiques. Cette proposition de loi, déposée par notre collègue députée Isabelle Santiago, présente aujourd'hui dans les tribunes à l'Assemblée nationale, après- il est vrai -un certain nombre de modifications et un travail avec la Chancellerie, a pour objectif de mieux protéger les enfants victimes et covictimes, directes ou indirectes, de ces violences. Ce texte est pour nous important, car il constitue un pas de plus vers la protection des enfants et prend place dans un continuum législatif qui, peu à peu, se consolide. À chaque fois, nous sommes au rendez-vous.

sur des victimes mineures, en insérant dans le code pénal de nouvelles infractions d'agressions sexuelles autonomes sur mineur de moins de 18 ans dans le cas de l'inceste.

Pour nous, la question de la protection des enfants victimes ou covictimes de violences intrafamiliales doit être comprise dans un ensemble plus large, qui prend en compte aussi la protection du parent victime et la question de l'emprise du parent violent sur la victime par l'instrumentalisation de l'enfant. Protéger l'enfant est primordial, mais c'est aussi une manière de protéger le parent victime, la plupart du temps la mère. Rappelons que le nombre de féminicides a augmenté de plus de 20 % lors des trois dernières années et que nous en sommes à 34, déjà, pour l'année 2023.

Nous souhaitons aussi que la loi précise que la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement doit être effective dans un délai maximal de six jours.

Hannah Arendt écrivait que le développement de l'enfant était la continuité du monde. L'enjeu de cette proposition de loi est de faire en sorte que les enfants ne soient pas tributaires d'un passé douloureux, marqué par la violence, responsable de traumas lourds. Les études et les statistiques sont glaçantes, sans équivoque : 60 % des enfants témoins de violence souffrent de stress post-traumatique ; 50 % des victimes de viol durant leur enfance ont fait une tentative de suicide.

Grâce à la mobilisation des mouvements et des associations féministes, les violences faites aux femmes et les féminicides ne sont plus considérés comme des drames passionnels, mais comme la résultante du système patriarcal qui gangrène nos sociétés.

Malheureusement, les enfants sont encore trop souvent des victimes collatérales, l'objet de chantages de la part de conjoints violents. Malgré les avancées législatives de 2019 et de 2020, les enfants ne sont toujours pas assez pris en considération. Mes chers collègues, non seulement nous devons protéger les enfants témoins de violences commises sur la personne de l'autre parent- dans la majorité des cas, la mère -, mais nous devons également faire en sorte que plus aucun enfant ne meure des suites de maltraitance. Aujourd'hui encore, un enfant meurt tous les cinq jours de maltraitance. Un an après l'adoption de la loi Taquet, nous considérons toujours que les moyens accordés à la protection de l'enfance sont insuffisants.

Pour ce qui me concerne, j'ai toujours considéré qu'un conjoint violent ne pouvait pas être un bon père, et je me réjouis que cette analyse soit de plus en plus largement partagée. La vulnérabilité des enfants nous commande de prévoir une protection stricte, sans concession. Nous regrettons par ailleurs que la présente proposition de loi ne traite pas de tous les cas de violence à l'encontre de l'enfant qui, quelle que soit leur forme, doivent être dénoncés. Ayons en tête que la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) nous oblige à protéger les enfants contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale. Mettons-nous réellement

tombe sous le coup de cet article. Il est impératif, dans l'intérêt de l'enfant, d'appliquer le principe de précaution. De même, il est grand temps d'en finir avec le prétendu syndrome d'aliénation parentale, trop souvent utilisé lors des conflits ou en cas de violences conjugales.

Enfin ! L'immuable lien entre parent et enfant peut enfin être considéré comme délétère lorsque le parent est violent. Que d'années perdues, que de vies abîmées, pour n'avoir pas su dissocier le père du mari, la femme de la mère, pour avoir nié l'évidence qu'un mari violent- car c'est souvent un mari -est un homme violent, un père violent Non, un enfant ne peut pas se construire de façon équilibrée dans un climat de violence. Même si cette dernière n'est exercée que sur la mère, elle constitue une violence pour l'enfant. d'une violence psychologique : l'enfant est pris dans un étau entre son père et sa mère, impuissant, inquiet pour sa propre sécurité face à un conflit qui, pour reprendre les termes du juge Édouard Durand, s'apparente à une scène de guerre ou à un attentat. que cela, car, dans une guerre ou après un attentat, l'enfant peut encore se réfugier dans les bras de l'un de ses parents. L'enfant n'a d'autre choix que de se taire, d'assister, impuissant, au délitement des piliers de son existence. Cette violence psychologique aura incontestablement des effets graves sur son développement, sur l'enfant qu'il est et sur l'adulte qu'il deviendra. Protéger l'enfant, c'est donc l'éloigner de cette violence, quitte à suspendre l'autorité parentale qui, rappelons-le, vise à protéger l'enfant, sa sécurité, sa santé et sa moralité, afin de garantir son éducation et de permettre son développement dans le respect respect dû à sa personne. L'autorité parentale est une responsabilité vis-à-vis de l'enfant, un devoir. Un parent violent n'est pas un bon parent. De nombreuses études montrent qu'un père violent se sert de ses enfants pour nuire à la mère ; car la victime est souvent la mère. Il l'utilise comme monnaie d'échange, y compris après la séparation. L'autorité parentale que peut exercer le parent violent, condamné, soumet l'enfant à une pression insidieuse, perverse, qui ne permet pas à l'enfant de se reconstruire et qui place la mère face à un danger permanent. Aujourd'hui, le bourreau dicte encore sa loi. Et que dire de la violence directe, de l'inceste ! À ce titre, je tiens à saluer tout particulièrement le travail et l'engagement de longue date sur ce sujet de notre rapporteure, Marie Mercier. La commission des lois a fait le choix d'autoriser la suspension en urgence, avant tout jugement, de l'exercice de l'autorité parentale d'un parent mis en cause pour les infractions les plus graves sur son enfant- crime, viol et agression sexuelle. Je comprends cette position équilibrée, qui tend à concilier présomption d'innocence et protection de l'enfant. Je souhaite cependant que nous puissions aller plus loin : plus que l'exercice de l'autorité, c'est bien l'autorité parentale en tant que telle qu'il faut suspendre, car le parent privé de l'exercice de cette autorité en reste néanmoins le titulaire. Ainsi, le parent poursuivi, mis en examen ou condamné pour des faits graves, conserve certains attributs fondamentaux de l'autorité parentale, comme le droit de surveillance de l'enfant. Il est important de corriger cette situation. Nous devons être plus ambitieux ! Pourquoi ne pas étendre le dispositif de l'article 1 aux atteintes sexuelles incestueuses ? Nous aurons l'occasion d'en rediscuter, madame la rapporteure. Je me félicite également du choix de la commission d'ériger en principe la suspension du droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour violences intrafamiliales. s'agit là encore d'une mesure de cohérence, qui aura pour effet d'acculturer les juges et de les inciter à porter un regard neuf sur ces dossiers complexes. En tant que présidente de la délégation aux droits des femmes et auteure de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, texte enrichi des apports du Parlement et complété par vos travaux, madame la rapporteure, je me félicite des avancées proposées aujourd'hui aujourd'hui par la commission des lois. Ce texte marque bien le début d'un changement profond dans notre manière d'appréhender les violences intrafamiliales et d'accompagner les victimes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi, qui aménage les conditions du retrait ou du maintien de l'autorité parentale et de son exercice en cas de violences intrafamiliales, est un texte attendu par de nombreuses associations.

L'autorité parentale ne peut pas se résumer à un droit sur l'enfant, car elle constitue un ensemble de droits et de devoirs qui, en principe, garantissent une protection à l'enfant dans le cadre de son éducation.

Cette réécriture assure la lisibilité du lien, désormais automatique, entre condamnation pour violences sur la personne de l'autre parent ou sur l'enfant et autorité parentale. Il s'agit d'une réelle avancée. De même, le texte initial prévoyait fort opportunément d'étendre la mesure de suspension automatique de l'autorité parentale, prévue à l'article 378-2 du code civil, aux violences provoquant une ITT de plus de huit jours sur l'autre parent, de viol ou aux agressions sexuelles incestueuses sur l'enfant. La commission a limité cette suspension aux cas les plus graves, considérant que, pour les autres cas, l'objectif visé était déjà satisfait par le droit. L'article 2, qui garantit l'individualisation des décisions des magistrats, pose le principe du retrait de l'autorité parentale avec, si je puis dire, une différenciation entre les obligations incombant aux magistrats en matière de prononcé de décision relative à l'autorité parentale ou son exercice. La possibilité pour le juge de maintenir l'autorité parentale ou son exercice sur décision spécialement motivée devra, quant à elle, permettre de prendre en compte les cas, même marginaux, de crimes commis à la suite de violences subies par l'un des deux parents. doute en tête, tout comme moi, la terrible histoire de Valérie Bacot. Avec force, les associations oeuvrant contre les violences faites aux femmes et, plus particulièrement, celles qui accompagnent les familles de victimes de féminicide, réclament une suspension automatique de l'autorité parentale jusqu'au procès. Cette demande se justifie par les situations dramatiques que vivent les enfants orphelins à la suite de féminicides, qui sont restés sous l'autorité parentale du parent survivant, voire pire, sous la menace de l'exercice du droit de visite. Ces cas sont rarissimes, mais en la matière- vous en conviendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues -, un cas c'est déjà trop Si je ne doute pas une seconde de la rigueur du travail des magistrats et de leur souci de l'intérêt de l'enfant, j'ai été étonnée, à la faveur des témoignages, par l'existence de disparités territoriales en matière de coordination.

L'article 2 élargit et précise les cas de délégation de l'autorité parentale. Il facilitera le quotidien des enfants recueillis et des familles les accueillant. Il existe en effet, hélas, des situations dans lesquelles l'autorité parentale peut devenir une arme entre les mains du parent. Les féminicides sont des drames que l'on n'anticipe pas.

Vous l'aurez compris, ce texte me semble contribuer à la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales. On ne peut que se féliciter de son enrichissement tout au long de son examen. La parole

Le Gouvernement n'a pas engagé la procédure accélérée sur ce texte, car il traite d'un sujet sensible, celui de la protection de l'enfance, qui requiert que toutes les précautions soient prises par le législateur.

notre assemblée. Elle s'inscrit dans la droite ligne de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Ce texte a introduit dans notre droit une distinction entre le retrait de l'autorité parentale et celui de l'exercice de l'autorité parentale. parentale. Il vise à élargir le mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale dans le cadre des procédures pénales, et à rendre plus systématique le prononcé du retrait de l'autorité parentale par les juridictions pénales en cas de crime commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent ou d'agression sexuelle incestueuse. Depuis 2016, le nombre de cas de violences intrafamiliales ne cesse d'augmenter. En 2019, 44 % des plaintes pour violences physiques et sexuelles enregistrées par les services de sécurité concernaient des violences commises au sein de la famille. Un pic a été atteint en 2020 en raison du confinement, mais la tendance à la hausse ne semble pas fléchir, comme le prouvent les chiffres enregistrés depuis 2021. La libération de la parole et l'encouragement à signaler toutes les formes de violences intrafamiliales ont sans aucun doute contribué à cette augmentation. Ces chiffres effrayants, derrière lesquels il convient de mettre des visages, nous obligent, en notre qualité de législateur, à agir : il s'agit pour nous d'enrayer ce phénomène. Je tiens à saluer le travail minutieux de réécriture effectué par notre rapporteur, Marie Mercier, qui maîtrise parfaitement ces mécanismes juridiques complexes, et qui a déjà beaucoup oeuvré sur le sujet des violences conjugales et intrafamiliales.

Le respect des principes généraux du droit, constitutionnels et conventionnels, que sont la présomption d'innocence, l'intervention nécessaire du juge appréciant l'intérêt de l'enfant, le droit à une vie familiale et privée normale, a très nécessairement guidé le travail de la commission des lois. que les amendements adoptés en commission ont permis de rationaliser et de mettre en cohérence le droit civil avec le droit pénal. Ainsi, à l'article 1, la commission réserve l'extension de la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement aux cas les plus graves, ceux de crime ou d'agression sexuelle incestueuse sur la personne de l'enfant. disposition permettra de suspendre en urgence, avant tout jugement, l'exercice de l'autorité parentale d'un parent mis en cause commission des infractions les plus graves sur son enfant, le temps qu'un juge se prononce.

L'article 2 prévoit de faire un principe du retrait total de l'autorité parentale en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant ou de crime sur l'autre parent. Enfin, l'article 3 contribuera à rendre plus cohérentes et effectives les mesures figurant dans cette proposition de loi.

et à mesure aux évolutions, parfois terrifiantes d'ailleurs, de notre société et de notre époque. Au fond, ce n'est pas le droit qui fait la société, mais la société qui fait le droit.

que, lorsqu'un enfant est en danger, la question de l'autorité parentale ou de son exercice ne se pose que dans un second temps. L'urgence est en effet, dans un premier temps, de mettre l'enfant à l'abri. Il existe alors plusieurs procédures possibles, bien souvent à la main du parquet qui joue un rôle central. En amont de toute poursuite, le parquet peut ordonner en urgence, et sans aucune procédure contradictoire, le placement provisoire de l'enfant, éventuellement chez l'autre parent, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours. Il peut aussi placer l'enfant dans un lieu de placement pour enfants en danger ; mais encore faut-il que des places soient disponibles. Le parquet peut également, à tous les stades de la procédure ou même en amont, requérir la délivrance d'une ordonnance de protection auprès du JAF, avec des mesures d'interdiction d'entrer en relation et de se rendre dans certains lieux, ou la suspension du droit de visite et d'hébergement. Enfin, dans le cadre d'une information judiciaire ou de procédures rapides de jugement, la personne poursuivie peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique. Là encore, peuvent être prononcées une interdiction d'entrer en contact et de paraître en certains lieux ou la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur. Mes chers collègues, il est nécessaire de garder à l'esprit que ces dispositifs se cumulent et que la mise à l'abri de l'enfant, à proprement parler, ne repose pas sur les articles 378-2 et 378 du code civil, dont nous discutons actuellement.

même non définitive, pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits. Je partage l'avis de Mme la rapporteure sur le point suivant : rien ne justifie de conditionner cette mesure au fait que l'enfant ait assisté aux violences. Selon le juge Édouard Durand, président de la Ciivise, l'ajout de cette condition de présence de l'enfant lors des faits permet de diviser par quatre ou cinq le nombre de dossiers à traiter. Or nous ne sommes pas ici pour réduire le nombre de dossiers aux dépens des victimes, mais pour renforcer la protection des enfants J'en profite donc pour remercier Mme la rapporteure d'avoir pris en considération l'amendement que j'avais déposé en commission et qui a été intégré au texte. Toutefois, il est fondamental de tenir compte des violences conjugales- et pas uniquement des crimes commis sur l'autre parent -comme motif de suspension de l'autorité parentale ou de son exercice. Nous devons consacrer la formule suivante : « Un parent violent ne peut pas être un bon parent. » C'est d'ailleurs l'un des objectifs de l'amendement que je défendrai dans quelques instants. rédigé, l'article 1 ne permet pas une prise en compte globale de la problématique des femmes victimes de violences conjugales et, intrinsèquement, des enfants victimes de violences intrafamiliales. Je suis saisi

ou condamné, même non définitivement, que ce soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, pour une agression sexuelle incestueuse, pour une atteinte sexuelle incestueuse, ou encore pour un crime commis sur la personne de son enfant, et ce jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales.

Il est primordial de préserver les enfants victimes durant le temps de l'enquête. Le doute doit profiter à la protection de l'enfant. Nous ne devons pas prendre le risque qu'un acte de nature pénale soit commis contre l'enfant pendant ce temps de latence. Mes chers collègues, la simple suspension de l'exercice de l'autorité parentale ne suffit pas à protéger efficacement les enfants victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. En effet, dans ce cas, l'autre parent a l'obligation de donner au parent poursuivi pour violences l'adresse du nouveau domicile

amendement vise à prévoir une suspension de plein droit de la titularité de l'autorité parentale, et non simplement de son exercice. La distinction entre exercice et titularité est primordiale. Un parent titulaire de l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant et conserve un droit de surveillance sur ce dernier. Le parent poursuivi, mis en examen ou condamné, conserve donc certains attributs fondamentaux de l'autorité parentale : nous souhaitons corriger cette situation. Nous estimons nécessaire de prendre en compte l'ensemble des violences sexuelles incestueuses commises à l'encontre d'un enfant, et voulons étendre les cas de retrait provisoire de plein droit de l'autorité parentale du parent poursuivi ou condamné au délit d'atteinte sexuelle incestueuse. La notion d'atteinte sexuelle permet d'englober un plus grand nombre de cas dans lesquels l'enfant est victime d'inceste et de lui assurer ainsi une meilleure protection. Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle non consentie.

à un nombre minimum de jours d'ITT ou à la présence de l'enfant. Il n'est pas question d'attendre que l'un des parents tue l'autre parent avant de mettre à l'abri le ou les enfants. La protection des enfants doit nous guider. L'amendement

et trop lourdes de conséquences pour les enfants qui en sont victimes pour ne pas conduire à la suspension de l'autorité parentale ainsi que des droits de visite et d'hébergement. Afin de faciliter le travail des juges et d'éviter une limitation excessive de la portée du texte sur ce point, nous proposons de rétablir la rédaction adoptée

à partir de huit jours d'ITT, ainsi que le crime ou l'agression sexuelle commis sur son enfant, sans délai maximal de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement. Nous considérons que ces deux dispositions constituent l'un des apports majeurs

une durée de six mois, même lorsque le parent est poursuivi par le ministère public, mis en examen ou condamné pour un crime commis sur l'autre parent, pour agression sexuelle incestueuse ou pour un crime

L'amendement vise également à intégrer, dans le champ de la procédure de suspension provisoire de plein droit, les atteintes sexuelles incestueuses, ce qui recouvre l'exhibition ou le visionnage de film pornographique en présence de l'enfant.

la mesure de suspension en étendant son champ à des délits, ce qui porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Compte tenu de son caractère automatique et de l'absence de toute intervention du juge, la commission a souhaité réserver la suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale aux seuls cas les plus graves- les crimes et les délits d'agression sexuelle incestueuse -et conserver les mêmes effets limités dans le temps qu'actuellement, soit une durée maximale de six mois jusqu'à la décision du JAF. De surcroît, la rédaction proposée pose de nombreuses difficultés techniques, car elle mélange les notions de suspension et de retrait. Les auteurs de l'amendement partent du principe que la suspension serait prononcée par un magistrat, alors qu'elle est de plein droit et s'opère automatiquement par simple effet de la loi en cas de poursuite par le ministère public, de mise en examen par le juge d'instruction ou de condamnation. Elle n'est donc pas formalisée par une décision qui pourrait acter un retrait

Par ailleurs, en cas de condamnation pour violences conjugales de nature délictuelle, selon les dispositions du décret du 23 novembre 2021, l'enfant témoin de ces violences est considéré comme une victime ; la juridiction pénale a donc l'obligation de se prononcer

tout en ajoutant un délai de six jours pour l'intervention de la suspension et en supprimant la condition relative à la présence de l'enfant pour ce qui concerne les violences conjugales. La commission a entendu limiter

de suspension particulier en cas de condamnation pour violences conjugales de nature délictueuse. Il appartient donc à la juridiction pénale de se prononcer, au moment de la condamnation, sur l'autorité parentale. C'est le sens de l'article 228-1 que nous avons introduit dans le code pénal au travers

ou de son exercice, ainsi que des droits de visite et d'hébergement. Le premier mécanisme, en cas de poursuite ou de condamnation du parent pour un crime commis sur l'autre parent ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur l'enfant, s'appliquerait jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, la décision de non-lieu du juge d'instruction ou la décision du juge pénal.

Je vous rejoins évidemment sur la nécessité de prévoir que le mécanisme de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que des droits de visite et d'hébergement s'applique aux crimes et aux agressions sexuelles incestueuses dont un enfant peut être victime. En revanche, il me paraît excessif de suspendre automatiquement- les adverbes ont beaucoup d'intérêt -la titularité même de l'autorité parentale alors qu'aucun juge n'a examiné la situation. Je

j'avais indiqué que celle-ci me semblait équilibrée. Pour des raisons constitutionnelles, il nous faut être prudents. Il est impératif de limiter le mécanisme de suspension de l'exercice de l'autorité parentale aux infractions les plus graves et aux violences conjugales entraînant un ITT de plus de huit jours, à condition qu'elles soient commises en présence de l'enfant.

déduis qu'elle peut être maintenue sur les autres enfants de la fratrie, ce qui, selon moi, pose un premier problème. Comment un père-

L'amendement n° 8 rectifié vise à rendre cette suspension automatique chaque fois qu'un parent est poursuivi pour un crime, un viol, une agression sexuelle ou la diffusion et l'enregistrement d'images à caractère pornographique d'un mineur de 16 ans.

Elle n'a pas non plus été envisagée par le législateur, puisque l'article 378 du code civil ne prend en considération que les crimes et délits commis sur l'enfant ou les crimes commis sur l'autre parent. Il me semble que ces dispositions élargiraient énormément le champ de la suspension automatique, au point d'encourir un grief d'atteinte à la proportionnalité. Plus on s'éloigne de l'enfant qui fait l'objet de l'autorité parentale, plus il faut se méfier des solutions automatiques. Gardons en tête que la situation de l'enfant doit être examinée, en fonction de son intérêt,

incestueuse commis sur la personne de son enfant » entraînerait le déclenchement de la suspension en cas d'infractions de natures extrêmement variées commises par l'auteur en dehors de son cercle familial.

la suspension de l'exercice de l'autorité parentale aurait lieu en cas de crime, quelle que soit la victime, qu'elle appartienne ou non au cercle familial de l'auteur. Une nouvelle fois, vous excluez du dispositif le mineur de 16 à 18 ans, qui ne serait plus protégé, même en cas de crime.

et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné pour des violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Une initiative législative visant à lutter contre les violences intrafamiliales et, qui plus est, à en protéger les enfants ne saurait faire l'économie de dispositions liant les violences conjugales à une suspension de l'exercice de l'autorité parentale.

précédent. J'insiste sur ce point : il est extrêmement important d'ajouter le délit d'atteinte sexuelle incestueuse à la liste des cas dans lesquels le parent condamné se voit retirer totalement l'autorité parentale.

son enfant ». Le groupe RDPI souscrit pleinement à cette proposition, qui participe d'une meilleure protection des enfants victimes de violences sexuelles. Or force est de constater que la rédaction adoptée par la commission des lois des lois ne garantit pas le caractère systématique du retrait de l'autorité parentale, le juge devant seulement se prononcer sur le sujet. Aussi, pour redonner sa pleine portée au dispositif, nous souhaitons que le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice soit systématiquement ordonné par le juge, sauf décision contraire spécialement motivée. Par ailleurs, dans un souci de clarté et de lisibilité, nous suggérons de fusionner les alinéas 4 et 5 afin de permettre au juge de retirer l'autorité parentale ou son exercice en cas de condamnation d'un parent

de la mesure. Ainsi, il a semblé plus juste à la commission de distinguer entre l'obligation de se prononcer et l'obligation de motiver spécialement une décision autre que celle d'un retrait total de

autre qu'une agression sexuelle incestueuse, peuvent ordonner le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice. Sur ce point, l'amendement est moins-disant que le texte de la commission, lequel impose aux juridictions, dans ce cas, de se prononcer

Le retrait automatique de la titularité de l'autorité parentale ou, à défaut, de son exercice nous semble problématique. Nous ne voyons pas pour quelle raison nous devrions craindre l'intervention du juge. Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

en supprimant la référence au droit de garde, lequel n'existe plus depuis 1987.

de prononcer un retrait de l'exercice de l'autorité parentale plutôt qu'un retrait de l'autorité parentale. Il semble donc nécessaire de conserver les deux visas. L'avis est défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

doit être supprimée, car cet article ne porte que sur le retrait de la titularité de l'autorité parentale dans le cadre civil, alors même que l'objet de l'article 2 en est d'instaurer un délai avant lequel il n'est pas possible de saisir le JAF pour demander la restitution de l'exercice de l'autorité parentale, retiré dans un cadre pénal, sur le fondement de l'article 378 du code civil. Je suis donc favorable à cet amendement.

Le code civil dispose que ce délai, d'une durée maximale de six mois, court jusqu'à la décision du juge. Charge alors au procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours.

ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Quant aux violences sur l'enfant, c'est une évidence : le rôle même du JAF

Par ailleurs, les violences conjugales sont évidemment un élément à considérer par le JAF au moment de prendre sa décision. L'article 373-2-11 du code civil prévoit expressément que celui-ci, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, tient compte

en cas de condamnation pour un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, commis par un parent sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent. Le lien enfant-parent ne doit pas être maintenu à tout prix et il est préférable que l'enfant soit préservé de tout contact avec celui qui s'en est pris à sa vie ou à celle de son autre parent. Préserver un tel lien serait contre-productif et toxique. On ne peut pas penser qu'un enfant puisse se reconstruire lorsqu'il est contraint de revoir son bourreau

à tous les crimes et délits commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent. Cette disposition offre une meilleure intelligibilité et favorise la cohérence entre code civil et code pénal. Hormis cette différence de structure, l'amendement n° 20 est satisfait par l'article 3 tel que rédigé par la commission.

est à Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous souhaitons que la juridiction de jugement puisse ordonner systématiquement le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour un viol une agression sexuelle incestueuse ou une atteinte sexuelle incestueuse commis contre un mineur par une personne titulaire de l'autorité parentale sur celui-ci. Comment concevoir qu'une marge d'appréciation demeure demeure au cas par cas dans de telles situations incestueuses ? Pour le bien de l'enfant, pour son avenir et sa reconstruction, il est fondamental que le retrait de l'autorité parentale soit automatique dans ces circonstances. Aucune raison ne saurait justifier le maintien de l'autorité

Cet article prévoit un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice, notamment lorsque le parent s'en est pris à son enfant dans les conditions qui ont été indiquées précédemment. Il doit en être ainsi, en particulier lorsque des actes incestueux ont été commis. Par la transgression de l'interdit fondamental de nos sociétés, de tels actes justifient un retrait définitif et automatique des attributs de l'autorité parentale. Retirer l'autorité parentale à celui qui s'affranchit des interdits sexuels

Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à

qui est concerné par une procédure portant sur l'autorité qui s'exerce sur lui doit être considéré comme une personne à part entière et, à ce titre, être systématiquement représenté par un avocat lui étant entièrement dédié.

Quel est l'avis de la commission ?

: La parole est à M. François Bonneau. Cet amendement vise à compléter les dispositions du code de procédure pénale afin de systématiser la suspension, par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des droits de visite et d'hébergement du parent mis en examen pour une infraction incestueuse.

Par cet amendement, nous souhaitons garantir le respect de l'enfant par l'écoute de sa parole. Nous pensons que chaque enfant doit être entendu dans sa singularité, et qu'aucune généralisation ne doit gommer

Il est précisé que la parole de l'enfant doit être recueillie sans aucun préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement. Quel est l'avis de la commission ?

la proposition de loi présentée par notre collègue Isabelle Santiago à l'Assemblée nationale. Nous sommes en effet très attachés à l'égalité entre les femmes et les hommes, et particulièrement révoltés contre toute toute manifestation de violence à l'égard des femmes. La persistance d'un système qui minimise les violences, néglige leurs conséquences et hésite à sanctionner les auteurs constitue une entrave à la liberté des femmes victimes et à l'instauration de cette égalité. Nous souhaitons corriger les failles de notre justice familiale et pénale, cette justice qui laisse parfois entendre qu'un mauvais mari pourrait être qu'un mauvais mari pourrait être un bon père. Cette justice qui néglige les conséquences des conflits perpétue le continuum des violences. Que vaut aux yeux de l'enfant la loi qui ne l'a pas protégé de la violence d'un parent ?

présidée par le juge Édouard Durand, estime dans son rapport que 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année en France, un nombre longtemps sous-estimé, voire négligé, en particulier en raison du tabou anthropologique dont ce crime fait l'objet. Plus largement, une personne sur dix est victime d'inceste dans son enfance, soit plus de 5 millions de femmes et d'hommes. Pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste votera cette proposition de loi visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales. Comme je l'indiquais dans mon propos liminaire, ce texte n'est pas une fin en soi ; il marque le début d'un changement profond de l'approche de notre société sur les violences intrafamiliales, prenant en compte que le parent violent n'est jamais un bon parent. Les débats et les propositions d'amendements issues de toutes les travées de notre assemblée attestent notre volonté collective d'améliorer le texte. La navette- je n'en doute pas -apportera des avancées nouvelles,

Elles apportent également aux collectivités des moyens et des outils nouveaux dans leur gestion quotidienne des déchets. Depuis ma prise de fonctions, je travaille pour que les collectivités disposent des moyens financiers suffisants pour rendre le traitement des déchets plus performant. C'est à ce titre que, pour 2023, le fonds vert alloue une enveloppe de 60 millions d'euros à la collecte et à la valorisation des biodéchets. En parallèle, 90 millions d'euros ont été ajoutés au fonds économie circulaire. suis enfin engagée à revoir les barèmes de soutien au regard de la crise énergétique que nous vivons et que les collectivités subissent de plein fouet. Notre politique de développement de l'économie circulaire fait figure d'exemple sur la scène européenne et internationale. Je souhaite Je souhaite que le texte que nous examinons aujourd'hui s'inscrive dans cette dynamique. Cette proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale posait un principe clair : donner les moyens à la filière papier-carton de gagner en performance environnementale la fusion des REP papier et emballages. Il avait aussi pour objectif de pérenniser, pour le secteur de la presse, la possibilité de contributions en nature, en prévoyant l'accès direct et majoritaire des collectivités à ce dispositif tout en restant exigeant sur l'ambition environnementale fixée par l'État dans Les filières REP sont les clés de voûte de notre système de financement et de gestion des déchets. Elles sont aussi à la base de notre système de prévention, de réparation, de réemploi et de propreté.

Au-delà de la cohérence et de la simplification recherchées, cette fusion permet également d'avoir une vision commune entre ces deux filières concernant l'écoconception, et partant, de gagner en performance environnementale. Par ailleurs, la filière papier connaît un changement d'équilibre économique. En seulement deux ans, l'activité de production de papier a diminué de 12 %, et cette trajectoire perdurera. Dans ce contexte, la fusion devra dans tous les cas avoir lieu tôt ou tard. En la votant dès à présent, nous prenons nos responsabilités quant à la pérennité de la filière. Cette fusion permettra de mieux partager les coûts structurels de gestion du bac jaune et du recyclage, et ainsi, d'améliorer l'assise et la visibilité financière de la filière.

Pour autant, et j'y tiens particulièrement, il n'est pas question d'exonérer un secteur de sa responsabilité environnementale et de minimiser le manque à gagner pour les collectivités. de ce texte, nous nous sommes donc tous interrogés sur la meilleure manière d'adapter le dispositif de responsabilité de la presse sans freiner l'ambition environnementale du secteur.

A également été ajouté le fait de quantifier chaque année les économies dégagées par cette mise à disposition gratuite d'encarts pour les collectivités. Ensuite, la lecture à l'Assemblée nationale a permis d'enrichir le texte de critères environnementaux demandés au secteur de la presse. Il a ainsi été que les encarts concernent, en plus du geste de tri et de l'économie circulaire, la préservation de la ressource en eau et la protection de la biodiversité. Par ailleurs, le texte a précisé que les exigences environnementales qui s'appliquent au secteur de la presse ne pourront pas être en dessous de celles que le secteur doit respecter jusqu'au 1 janvier 2023. commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la semaine dernière, a fait le choix de ne pas retenir cette disposition. J'en prends acte. J'émets néanmoins des réserves sur la solidité juridique du dispositif prévu dans le texte que nous allons examiner

En second lieu, les bonus imaginés pour la mise à disposition gratuite d'encarts d'information devront bien être compensés par l'augmentation des écocontributions d'autres personnes. L'idée du dispositif proposé par la commission du Sénat serait de faire supporter cette compensation par le seul secteur de l'emballage. Cette piste soulève toutefois une interrogation sur l'équité de ce dispositif. Il me semble donc juridiquement fragile. D'un point de vue écologique ensuite, le dispositif adopté en commission revient à ouvrir à tous les acteurs de l'emballage et des papiers la possibilité de bénéficier d'un bonus financier s'ils mettent à disposition gratuitement des encarts. Mais pour ajouter des encarts d'information équivalents à ceux que peut proposer la presse, il faudrait ajouter du suremballage. En d'autres termes, le dispositif adopté en commission incite les producteurs à ajouter encore plus d'emballages. Madame la rapporteure, vous conviendrez que ce n'est pas l'esprit de la loi Agec, à laquelle nous sommes tous attachés. C'est même à l'opposé du combat que nous menons et que vous menez aussi, et à l'opposé de ce que nous demandent les citoyens et les responsables politiques.

Il me semble primordial que le dispositif qui sera voté à l'issue de la navette parlementaire intègre cette exigence. Pour conclure sur ce point, le Gouvernement maintiendra son ambition dans le déploiement de toutes les filières REP de la loi Agec et il n'y aura aucune remise en cause de ces filières. Certaines sont en cours de mise en oeuvre, dès cette année, comme la filière REP bâtiment, celle des véhicules hors d'usage, celle des pneumatiques ou encore celle des emballages de la restauration. D'autres viendront plus tard comme la filière des textiles sanitaires à usage unique en 2024 ou encore la filière REP des déchets d'emballages industriels et commerciaux en 2025. La mise en oeuvre de ces filières REP est une attente forte des collectivités. Sachez qu'elle est entendue et qu'elle guide mon action au quotidien. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, pour celles et ceux qui étaient présents dans cet hémicycle à l'automne 2019 pour débattre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, l'échange que nous aurons ce jour aura, à l'évidence, un goût de déjà-vu. En effet, il y a quatre ans environ, nous avions dans cet hémicycle largement complété la copie proposée par le Gouvernement, afin notamment de renforcer la responsabilité élargie des producteurs, une application du principe pollueur-payeur qui permet de transférer le coût de la prévention et la gestion des déchets aux producteurs. Pour les filières couvertes par le service public de gestion des déchets géré par les collectivités territoriales, la responsabilité élargie des producteurs se traduit par un soutien financier des producteurs aux collectivités territoriales des contributions financières transitant par un éco-organisme. Il y a quatre ans, le de la loi Agec était très clair. Oui, les collectivités territoriales doivent améliorer la prévention et la gestion des déchets, en modernisant leurs centres de tri, en mettant en place la collecte séparée des biodéchets ou encore en développant la collecte hors foyer ; mais ces politiques ont un coût. La loi Agec prévoyait donc de renforcer la responsabilité élargie des producteurs pour que l'amélioration de notre politique d'économie circulaire pèse non pas exclusivement sur le contribuable local, en aval, mais aussi sur le producteur, en amont. Nous avons donc créé de nouvelles REP, par exemple sur les produits et matériaux de construction ou sur les articles de bricolage, de jardinage et de sport. Nous avons aussi étendu des REP existantes : une REP emballages professionnels a par exemple été créée pour compléter la REP emballages ménagers. Le sens de l'Histoire était donc celui de la montée en puissance des filières REP, concomitante de celle du service public de gestion des déchets. Les choses se sont depuis quelque peu déréglées, car la mise en place ou l'extension des REP a pris du retard de manière importante dans le cas de la REP bâtiment, pourtant très attendue dans nos territoires pour lutter contre les dépôts sauvages. Les contraintes sur les collectivités territoriales n'ont, quant à elles, pas été reportées.

C'est dans ce contexte qu'est arrivée la proposition de loi dont nous débattons ce soir. N'ayons pas peur des mots : ce texte est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour nos collectivités territoriales. pas celui qui est relatif à la fusion des filières REP emballages ménagers et papier, à laquelle notre commission est favorable et qui ne constitue pas le coeur du texte dont nous sommes saisis saisis ; il porte sur la sortie de la presse de la REP. Disons-le clairement : exclure la presse de la REP, comme le prévoyait la proposition de loi initiale, revient à faire payer, une fois de plus, les collectivités territoriales. Je rappelle que tout ce qui n'est pas pris en charge par les metteurs sur le marché doit être financé par les contribuables locaux. J'entends déjà ceux qui estiment que le manque à gagner pour le service public de gestion des déchets est limité- une vingtaine de millions d'euros -et pourrait être facilement absorbé par les collectivités. Je répondrai que sortir la presse de la REP pourrait constituer un dangereux précédent susceptible d'affaiblir l'ensemble des REP et, partant, le financement du service public de gestion des déchets. Ce serait en effet la première fois dans l'histoire de ce système, né en France dans les années 1990 et ayant essaimé partout en Europe, qu'un gisement serait retiré de la REP. D'autres secteurs pourraient à l'exemple de ce premier régime d'exception demander des aménagements et des exonérations pour l'avenir, au détriment des collectivités territoriales et de la protection de l'environnement. Nous ne pouvons pas accepter une telle régression environnementale et une telle atteinte au service public de gestion des déchets géré par nos collectivités territoriales. Cela étant dit, nous nous devons d'apporter une réponse au secteur de la presse, qui est actuellement en grande difficulté. Je le dis ici avec fermeté, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire avec mes collègues sénateurs de la commission de la culture, en premier lieu desquels le président Lafon et Michel Laugier, avec qui j'ai beaucoup échangé lors de mes travaux préparatoires. Je salue à cet égard le travail de Michel Laugier, dont le récent rapport a mis en exergue les difficultés conjoncturelles et structurelles auxquelles fait face la presse, notamment notre presse quotidienne régionale : doublement du prix du papier en un an, augmentation des coûts de l'énergie et diminution structurelle des ventes de la presse papier de 5 % par an. Nous nous devons d'aider la presse, cela est certain. Fallait-il, pour autant, le faire aux dépens des collectivités territoriales, au risque de fragiliser le bel édifice que constitue la loi Agec, matrice de notre politique d'économie circulaire ? Bien évidemment, Le Gouvernement avait d'autres options pour concilier protection du service public de gestion des déchets et préservation du secteur de la presse. Il n'a tout simplement pas voulu les étudier. La première option était que l'État prenne sa responsabilité en aidant le secteur de la presse à payer son écocontribution à compter du 1 janvier 2023. Il ne l'a pas fait. La seconde option, c'est celle que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adoptée la semaine passée. Le texte issu des travaux de notre commission maintient en effet la presse dans le champ de la REP, mais en permettant de moduler les contributions financières de la filière REP pour les produits contribuant à une information du public d'intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts, sous réserve de respecter des critères de performance environnementale fixés par décret. Cette modulation des contributions sous forme de prime pourra pleinement bénéficier aux publications de presse. Les avantages de cette proposition sont nombreux. Elle préserve l'intégrité de la REP en maintenant la presse en son sein. Elle est financièrement neutre pour le service public de gestion des déchets, car les primes versées devront être compensées par la filière REP. Elle offre enfin des garanties environnementales, en conditionnant l'octroi des primes à l'atteinte de critères de performance environnementale. Elle répond enfin clairement aux préoccupations du secteur de la presse, qui pourra continuer à utiliser le système existant des encarts. Cette option avait d'ailleurs été envisagée par les services ministériels au cours des travaux préparatoires à la loi Agec que j'avais menés il y a quatre ans. Cette proposition me semble plus robuste juridiquement que la convention de partenariat hors REP qui était proposée dans le texte initial. Contrairement à la proposition faite par les députés, nous nous appuyons en effet sur un outil bien connu, appliqué dans l'ensemble des filières REP : la modulation des écocontributions. Le législateur peut tout à fait créer des critères d'écomodulation qui ne sont pas spécifiquement prévus par le droit européen et qui n'ont pas trait à l'écoconception du produit : c'est par exemple le choix que nous avions fait dans la loi Agec, en créant un critère d'écomodulation pour les produits ayant une visée publicitaire ou promotionnelle. Je suis consciente que ce choix est moins confortable qui est proposé dans le texte initial, car il devra en assumer les conséquences et mettre en oeuvre les modulations proposées au sein de la filière REP. Il eût sans doute été plus confortable pour lui de laisser le législateur assumer seul la responsabilité de faire payer les collectivités territoriales. Vous l'aurez compris, ma priorité est d'abord de préserver les filières REP pour protéger le service public de gestion des déchets et nos collectivités territoriales. Elle est ensuite d'aider la presse, en lui apportant une réponse proportionnée pour faire face aux difficultés auxquelles elle fait face.